avis n° 122). Mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s'effectuera depuis les terminaux de vote. Je vous invite donc à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l'insérant

Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.

sociale (PLFSS) est avant tout un vote d'approbation ou de non-approbation des grandes orientations de la politique gouvernementale en matière d'action sociale. Je ferai trois remarques d'ordre général sur ces problématiques.

C'est un texte de fin de mandat sans relief. Concernant sa trajectoire financière, les inquiétudes que nous avions exprimées face à votre choix de maintenir sans perspectives la sécurité sociale en déficit n'ont reçu aucune réponse claire du Gouvernement. Et si notre amendement sur les recettes, concernant la taxe sur les valeurs mobilières, place la cinquième branche à l'équilibre, il a été adopté contre votre avis. En 2017, votre majorité a trouvé les comptes de la sécurité sociale proches de l'équilibre, après des années d'amélioration continue. Vous partirez en les laissant dégradés, dégradation qui a débuté dès 2018, car personne ne vous reprochera, bien sûr, les dépenses liées à la pandémie, mais vous partirez surtout sans avoir tracé un chemin de redressement. Si cette situation était le prix de changements structurels tirant les leçons de la pandémie, ce pourrait être le signe d'investissements utiles. Mais il n'en est rien. Dans notre explication de vote l'année dernière, nous disions déjà que le temps des crises doit être celui du changement. Or qu'observons-nous à l'issue de l'examen du PLFSS pour 2022 ? que le texte ne porte pas les changements dont notre système de sécurité sociale aurait besoin, ni sur la santé ni sur l'autonomie. Des mesures sont positives, bien sûr, comme dans tout PLFSS. Je pense au dispositif

Si ce PLFSS n'a pu être l'occasion de traduire financièrement de nouvelles organisations en santé, c'est bien parce que vous vous êtes privés d'une loi, vous contentant d'un texte printanier sans portée, dont certaines dispositions doivent déjà être repoussées. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvés à modifier les rapports entre les professions de santé dans la précipitation des amendements déposés après que l'examen du texte eut débuté au Parlement. Cette méthode brutale, irrespectueuse des négociations professionnelles et conventionnelles, a braqué. Elle a créé des conflits entre des professionnels qui doivent au contraire, alors que la ressource est parfois rare, mieux travailler ensemble au bénéfice des patients. Il en résulte que le Gouvernement oppose les soignants entre eux en alimentant un débat qui se réduirait à des conservatismes et à du « lobbyisme » alors que la question est celle de la cohérence de parcours de soins coordonnés et d'une optimisation du temps des différentes professions du soin, ainsi que du respect dû à chacun. S'agissant de la cinquième branche, dont nous approuvons la création, elle reste elle aussi dans un déficit de cadre, d'objectifs et de dispositifs, qui démontre malheureusement une absence de volonté politique. L'abandon de la loi Autonomie est un renoncement inacceptable. Devons-nous nous satisfaire que le ministre des comptes publics ait expliqué que la cinquième branche serait à l'équilibre en 2030 alors même qu'il n'en connaît pas plus que nous le contenu ? Doit-on en conclure, monsieur le ministre, que le Gouvernement intègre le renoncement à toute ambition forte en la matière ?

Car, bien sûr, on ne peut réformer notre système de retraites au détour du PLFSS, d'autant que votre projet est d'ajouter encore des conditions à l'obtention d'une pension complète alors même que nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à ne plus être en activité à l'heure du départ. En quelque sorte, vous proposez une réforme pour 50 % de la population, alors que la dégradation des conditions de travail, dans de nombreux secteurs, rend cette perspective socialement injuste et souvent physiquement irréaliste.

Ce vote contre, je le dédie à l'hôpital public, qui mérite beaucoup mieux. Il est en grande difficulté alors qu'il constitue un service public essentiel et précieux. La crise de la covid a révélé et amplifié le manque de soignants et le découragement de celles et de ceux qui exercent ces métiers. Monsieur le ministre, vous avez affirmé payer « trente ans d'incurie je vous souhaite, quand, dans quelques mois, vos fonctions prendront fin, de poser sur la situation un regard plus équilibré. Le Gouvernement aime à comparer ses actions avec celles de ses prédécesseurs, pensant trouver Vous regarderez bientôt vos actions en constatant que les Français et les soignants sont nombreux à en être désolés ! La parole

c'est désormais un lieu commun, et pourtant il est difficile cette année d'y échapper : le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est un texte ambitieux qui s'inscrit dans un contexte sanitaire et économique rare. C'est en effet le deuxième texte depuis le début de la pandémie de la covid-19. Il consacre, à ce titre, des dépenses exceptionnelles pour répondre à la crise sanitaire. Près de 5 milliards d'euros sont ainsi prévus en 2022 pour satisfaire la demande de tests et de vaccins, notamment. en baisse par rapport à 2020 et à 2021 compte tenu de perspectives heureusement plus favorables. Ce PLFSS prévoit,

ce texte l'est également par les mesures qu'il vise à prévoir en faveur de notre système de santé, conformément aux engagements du Ségur, notamment en matière de revalorisations salariales pour les personnels des établissements de santé, des Ehpad et du secteur médico-social. Il permettra surtout de poursuivre la réforme de l'autonomie initiée l'année dernière avec la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, en instituant un tarif plancher de 22 euros pour les services à domicile et en renforçant la présence médicale au sein des Ehpad. Citons également l'octroi automatique de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse, le remboursement de la contraception pour les femmes de moins de vingt-six ans ou la généralisation de la télésurveillance. Nous nous félicitons de l'état d'esprit qui a guidé les travaux du Sénat ces derniers jours et des avancées concrètes qui ont été enregistrées. Nous nous réjouissons, en particulier, que plusieurs de nos amendements aient été adoptés. Ils concernent l'interopérabilité de la télésurveillance et des dispositifs médicaux, le report de la réforme de financement des soins de suite et de réadaptation, les SSR, ou l'inclusion de territoires ultramarins dans les expérimentations consacrées aux masseurs-kinésithérapeutes, aux orthophonistes et aux infirmiers en pratique avancée. À l'inverse, nous déplorons que le Sénat ait décidé la suppression des mesures relatives à l'isolement et à la contention, de la carte professionnelle dans le secteur du domicile, de la protection sociale complémentaire des travailleurs de plateformes ou encore de la possibilité de report pour la contractualisation dans le cadre de la reprise de dettes des hôpitaux. Surtout, le Sénat a souhaité introduire au terme de notre examen un amendement relatif à la réforme des retraites, amendement qui ne saurait trouver sa place dans ce texte et qui, à lui seul, pourrait expliquer que nous nous abstenions Permettez-moi, mes chers collègues, puisque l'occasion m'en est donnée, de m'arrêter quelques instants sur la situation de nos comptes sociaux, c'est-à-dire sur la soutenabilité et la pérennité de notre modèle de protection sociale. Le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale pour 2021 a confirmé que la crise sanitaire a imputé fortement l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, en particulier ceux de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse Elles ont subi en 2020 un déficit de 39,7 milliards d'euros, et connaîtront en 2021 un déficit proche de 34 milliards d'euros. Nous pourrions, bien sûr, passer des heures à débattre des options, des orientations et des préconisations. Les chiffres, en revanche, sont têtus Alors, oui ! face à cela, nous ne devons pas faire l'économie de vrais débats, de belles querelles sur les vraies solutions à retenir pour préserver notre système. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées lors de nos précédents débats, notamment à l'occasion de l'examen des PLFSS, ou sous la forme de recommandations de la Cour des comptes. Comment maîtriser, si ce n'est réduire, les dépenses de l'assurance maladie sans modifier le niveau de prise en charge sanitaire de nos concitoyens, dépenses qui augmentent mécaniquement plus vite que les recettes au fil des années ? La référence de l'exécution de l'année 2019 à une projection à 2025- abstraction faite de la crise sanitaire -en est une illustration Les dépenses ont augmenté de 10 % quand les recettes peinent à atteindre les 4 % pour la seule branche maladie. Les principaux postes du PLFSS, branche maladie et vieillesse, sont tous les deux déficitaires, quelles que soient les prévisions à court et à moyen termes. La constitution de l'enveloppe Ondam, qui est à 84 % essentiellement consacrée aux dépenses de ville et aux dépenses des établissements de santé, ne peut échapper à une réorganisation en profondeur en 2018, les dépenses de pathologies et des traitements chroniques ont représenté 61 % de la dépense remboursée par l'assurance maladie, soit 102 milliards d'euros sur un total de 167 milliards. Nous n'échapperons pas également à des actions soutenues pour limiter les actes inutiles, voire à une nouvelle approche qui orientera, à moyen terme, notre modèle vers davantage de prévention et un réarmement de notre recherche. Nous devons prendre acte de l'échec de notre gouvernance déconcentrée, mais insuffisamment décentralisée. Des outils de la territorialisation ont en effet été créés, mais n'ont pas encore apporté la lisibilité nécessaire pour nos concitoyens ni produit l'efficacité attendue. Je pense, notamment, aux groupements hospitaliers de territoire (GHT), aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et aux conseils territoriaux de santé (CTS). Il nous faut également approfondir une approche fondée sur les bassins de vie sanitaires, qui fait chaque année ses preuves

les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement devrait nous permettre de définir avec davantage d'acuité les objectifs prioritaires en matière santé ainsi que la stratégie d'investissement.

Je vous remercie

nous avons examiné la semaine dernière le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Les débats ont été l'occasion d'évoquer des sujets importants visant à renforcer l'accès aux soins et aux droits sociaux des Français. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires a abordé cet exercice de façon pragmatique, en apportant autant d'idées nouvelles et de propositions d'amélioration que le couperet des articles sur la recevabilité des amendements le permet. L'Ondam a été revalorisé de 1,7 milliard d'euros en 2021 afin de compenser les surcoûts engendrés par la crise sanitaire, notamment pour les hôpitaux. Avec les dernières estimations macroéconomiques, le déficit des comptes sociaux s'établit à 20,4 milliards d'euros en 2022, soit 1,2 milliard de moins que les prévisions. Nous saluons l'extension des revalorisations salariales du Ségur de la santé à 20 000 professionnels du secteur du handicap exerçant au sein d'établissements financés par les départements. La juste revalorisation des métiers du secteur médico-social est essentielle pour favoriser l'attractivité des métiers et préserver la qualité des soins dispensés. Nous sommes favorables au doublement de la contribution exceptionnelle des complémentaires santé, qui refusent de s'engager à modérer leur hausse tarifaire, en dépit des économies réalisées durant la crise, chiffrées à 2,2 milliards d'euros. La question de la juste répartition des compétences entre sécurité sociale et complémentaires santé se pose réellement, sachant que les frais de gestion des mutuelles sont particulièrement élevés, avec 7,6 milliards d'euros de dépenses chaque année. Les sénateurs de notre groupe avaient défendu en 2019 un amendement présenté par Daniel Chasseing visant à prévoir un stage dans un désert médical pour les internes en dernière année de médecine. En complément de ce dispositif, nous avons défendu plusieurs amendements, adoptés la semaine dernière, pour faciliter l'accès aux soins dans les déserts médicaux. au dispositif incitatif visant à instaurer des zones franches médicales dans lesquelles les médecins pourraient bénéficier d'exonérations de cotisations sociales. au dispositif plus contraignant visant à conditionner le conventionnement par l'assurance maladie des médecins à l'exercice au moins pendant six mois dans des zones sous-dotées en médecins. L'accès aux soins pour tous, en tout point du territoire, est notre priorité et l'enjeu des années à venir. Dans de nombreuses communes rurales, les médecins retraités ne trouvent aucun remplaçant pour reprendre leur cabinet et garantir le suivi médical des habitants. Si cette situation n'est pas nouvelle, la progression des déserts médicaux en France est préoccupante, nous devons apporter des solutions d'urgence et de long terme pour y remédier. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons défendu le maintien de l'article 40 sur l'accès direct des patients aux orthoptistes pour favoriser l'accès à la santé visuelle, tout en proposant de renforcer le cadre dans lequel se déroulent ces consultations. Nous avons également voté en faveur du remboursement de consultations chez un psychologue agréé. En lien avec l'entretien postnatal précoce instauré à l'article 44 , il serait intéressant de prévoir un accompagnement particulier des jeunes parents à risque de dépression post-partum : 30 % des mères sont concernées, mais aussi 18 % des pères d'après les récentes études. Nous avons soutenu l'extension de la gratuité d'accès à la contraception pour les jeunes femmes de moins de vingt-six ans, tout en soulignant qu'il faudrait étendre cette mesure aux jeunes hommes. Nous saluons l'adoption de l'article 49 visant à faciliter le versement des pensions alimentaires. Cette mesure devrait améliorer la situation financière des familles monoparentales, soit actuellement une famille sur quatre, dont une majorité de mères célibataires. Le principal défaut de ce texte est l'insuffisance de financement en direction des Ehpad, dont le taux d'encadrement en personnel soignant reste bien en deçà de l'acceptable au regard du degré de dépendance des pensionnaires et de leurs besoins d'accompagnement. Les sous-effectifs récurrents en personnel soignant engendrent une forte dégradation des conditions de travail et augmentent les risques de maltraitance. Nous saluons néanmoins l'adoption de l'amendement de Daniel Chasseing visant à ouvrir vers l'extérieur les pôles d'activité et de soins adaptés pour favoriser l'accès à la santé mentale de nos aînés vivant à domicile. Notre groupe est favorable au report de l'âge d'ouverture des droits à la retraite de 62 à 64 ans, mais nous souhaitons que cette mesure fasse l'objet d'un texte à part entière. Le principe de réalité exige une augmentation progressive de la durée d'activité des Français. Pour cela, nous devons actionner trois leviers : la prévention des maladies chroniques, la formation tout au long de la vie et des conditions de travail adaptées. Nous n'avons pas voté en faveur de la suppression de l'article 5 relatif à la reprise d'une partie de la dette hospitalière par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). Nous n'avons pas non plus soutenu la suppression de la trajectoire financière des comptes sociaux pour les quatre années à venir. Si l'annexe B présente une trajectoire peu optimiste pour les finances sociales, cette dernière traduit les effets imprévisibles de la crise sanitaire. Il nous paraît difficilement acceptable d'adopter un projet de loi de financement de la sécurité sociale dépourvu de sa dimension pluriannuelle. Le nécessaire retour à l'équilibre des comptes sociaux ne doit pas se réaliser au détriment du financement des hôpitaux et du secteur médico-social. Au regard de ces éléments, la majorité des sénateurs de notre groupe a fait le choix de s'abstenir.

Arrêtons-nous un moment sur ce montant et sur ce qu'il dit de notre protection sociale. Il traduit tout d'abord l'effort consenti dans la crise pour protéger les Français. Le système de santé, soumis à de fortes tensions, a tenu bon et pris en charge des flux de patients inédits. L'État a financé très largement les tests, les vaccins et les outils de réponse à l'épidémie. Au-delà, il a préservé, ainsi que l'Insee vient de le confirmer, le pouvoir d'achat des actifs des effets potentiellement dévastateurs des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus. virus. Au-delà de ce rôle de « stabilisateur automatique », traditionnel en période de basses eaux économiques, ce déficit traduit aussi des déséquilibres plus structurels qui interrogent plus profondément notre modèle social. Ce déséquilibre, en premier lieu, est celui de l'assurance maladie. Il est sans aucun doute le plus difficile à régler tant il imbrique un nombre d'acteurs et de problématiques complexes. Nous pourrions faire le constat simple d'un manque de recettes devant des besoins croissants, liés au vieillissement, au développement des pathologies chroniques ou encore à l'innovation thérapeutique.

en matière d'accès aux soins, qu'elles soient sociales ou territoriales, sont criantes, au point de devenir une préoccupation de premier rang pour les Français. L'hôpital, devenu le premier point d'entrée de notre système de soins et le réceptacle de ces dysfonctionnements, semble craquer de toutes parts.

L'assurance maladie, dont le tableau clinique est inquiétant, exigera donc davantage qu'un surcroît de recettes- d'ailleurs, nous n'en disposons pas. Les termes du débat sont certainement plus simples quoique cette simplicité ne s'attache pas à la mise en oeuvre des mesures nécessaires, dans un pays où l'attachement à partir à la retraite assez tôt est important. Devant l'équation démographique

Là encore, le chantier est d'importance. Rendons-nous à l'évidence : dans un système par répartition, où les actifs financent le revenu des retraités avec une croissance faible, un nombre réduit d'actifs ne pourra soutenir la charge d'un nombre croissant de retraités sans aucun changement.

Le vieillissement de la population est avéré ; le levier de la prévention de la perte d'autonomie est insuffisamment actionné pour infléchir cette tendance. Pour y faire face, la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée, sur le rapport de nos collègues Bernard Bonne et Michelle Meunier, pour une assurance couvrant ce nouveau risque, souscrite le plus tôt possible afin de limiter le montant des primes. La perte d'autonomie est un vrai risque assurantiel, bien qu'elle ne touche pas 100 % d'une classe d'âge et qu'elle porte sur une durée relativement circonscrite. Faute d'assurer son financement, la nouvelle branche Autonomie, d'ores et déjà en déficit, reste une promesse non tenue. La définition d'un cadre à la gouvernance encore imprécise, notamment pour ce qui concerne le rôle des départements, ne peut suffire à répondre au défi de la prise en charge digne des personnes âgées de ce pays. Nous connaissons l'attente et les besoins qui s'expriment. Ils sont immenses, y compris du côté des personnes qui travaillent dans ces secteurs- ils ont besoin de motivation, de reconnaissance, de professionnalisation des compétences. Or rien ne vient y répondre dans l'immédiat.

La crise de 2008 avait été suivie de tentatives pour réguler les dépenses, puis d'une véritable austérité fiscale. Le présent texte ne dit rien des choix qui seront faits : c'est une source d'inquiétude pour l'avenir, qui nous a conduits à rejeter la trajectoire pluriannuelle. lors, nous avons voulu exposer les nôtres. Au-delà de ces questions de fond, nous appelons au respect des prérogatives du Parlement, dont le rôle éminent reste bien de consentir à la dépense.

d'en finir avec les amendements de dernière minute, qui ne sont pas de bonnes surprises, et de cesser de gaver un texte déjà obèse d'articles additionnels dépourvus de tout lien avec ses enjeux financiers. Rappelons, ici, notre opposition constante à l'inscription dans ce texte de la reprise par la Cades de la dette des hôpitaux.

que la Constitution leur confie. Sous le bénéfice de ces observations, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, tel qu'issu des travaux du Sénat. La parole est à Mme Raymonde

déstabilisant des filières entières par un mouvement dramatique de démissions ou de transferts de personnel, au détriment de secteurs déjà durement marqués par un grave déficit d'attractivité.

Nous ne pouvons que nous en réjouir et lui suggérer, à la faveur d'un prochain déplacement, de tenir compte d'autres professionnels exclus des différents dispositifs de revalorisation salariale du Ségur, tels que les psychologues des établissements publics de santé,

des mesures de restructuration brutales de l'offre. Vous dites y renoncer cette année, après avoir indirectement reconnu qu'elles pèsent et continueront de peser sur l'hôpital en crise. L'hôpital public, sinistré par cette politique de sous-financement, a besoin de rompre avec cette austérité. Dès lors, il nous est impossible de nous réjouir des avancées, d'autant que l'hôpital n'a pas vu tous les coûts du Ségur compensés et ne dispose pas encore d'une vision pluriannuelle lui permettant de se relever par des projections à moyen terme. Le même constat vaut pour les mesures positives de la branche autonomie : les prévisions jusqu'en 2025 semblent résumer l'ambition et valoir solde de tout compte, sans autres ressources d'ampleur.

Ainsi, aucun effort n'est demandé à ceux qui sortent gagnants de la crise sanitaire. En revanche, on surtaxe les complémentaires santé, qui font pourtant face aux effets de rattrapage des soins au premier semestre 2021, conduisant au risque de déséquilibres techniques la

En parallèle, aucune mesure sociale d'envergure ne permet de lutter contre l'intensification de la pauvreté, notamment parmi les jeunes et les travailleurs précaires, par l'ouverture à des revenus minimums garantis. Nous regrettons la suppression de l'article relatif à la contention et à l'isolement.

Nous nous sommes réjouis de l'indemnisation des victimes exposées aux pesticides, en portant des points d'attention. Cependant, nous regrettons le retard pris pour l'indemnisation des victimes du chlordécone.

J'en prends pour exemple l'amendement que nous défendions pour que les services domiciliaires puissent candidater de la même façon que les Ehpad lors de la création des centres de ressources territoriaux. Il a été déclaré irrecevable alors que son adoption n'aurait eu aucun impact sur le nombre de centres ouverts par la tutelle, donc aucun impact financier en soi.

En conclusion, prenant acte des avancées de ce texte, mais condamnant l'absence de volonté politique de trouver les ressources nécessaires au redressement durable de l'hôpital, à la lutte contre l'intensification de la pauvreté et à la couverture durable du risque autonomie, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre le projet

Le débat l'a mis plusieurs fois en évidence : ce PLFSS ne cherche pas à trouver de nouveaux financements, comme nous vous le proposons. Pis, les exonérations de cotisations deviennent la règle ! Votre entêtement fait perdre la modique somme de 150 milliards d'euros par an à l'État et à la sécurité sociale. Vous vous inscrivez dans la lignée de vos prédécesseurs. La remise en cause de la cotisation comme fondement de la sécurité sociale, par la création de la CSG,

est la seule création de richesses sans capital. La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget des contribuables pour la financer serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières. » C'est pourtant ce que que fait le Gouvernement ! Et tout cela a des répercussions : face aux conditions de travail dégradées, aux fermetures de lits, les départs se succèdent à l'hôpital. Tous nos territoires sont touchés, mes chers collègues. Alors que le service des urgences du centre hospitalier de Laval a fermé ses portes quelques nuits, il y a peu, les soignants dénoncent un manque de médecins endémique et une logique de restrictions budgétaires continues poussant cet

pour protester contre votre politique. Vous voyez bien, monsieur le ministre, que l'insatisfaction et la colère sont grandes dans le monde de la santé et le secteur médico-social. De plus, on ne peut être qu'inquiets face à la pandémie, qui regagne du terrain. Du côté de l'accompagnement de nos aînés, le ciel n'est pas davantage dégagé. La réforme de l'autonomie promise est enterrée ; pas de grand service public, pas de financement à la hauteur dans le cadre de l'assurance maladie. À la place, vous proposez une cinquième branche qui assure ses financements à coups de CSG et de recettes

avancées demeurent limitées ; elles ne suffisent pas à modifier la philosophie globale de ce budget de la sécurité sociale, qui met des rustines sur les difficultés d'accès aux soins. Nous sommes favorables à une reconnaissance des compétences des professions

que nous repensions de fond en comble l'organisation de notre système de santé et de protection sociale. Elle appelait à rompre, une bonne fois pour toutes, avec les choix qui, depuis des décennies, tuent à petit feu notre système de santé et de protection sociale. Ce n'est malheureusement pas la voie que vous avez empruntée, monsieur le ministre, pas plus d'ailleurs que la majorité sénatoriale : sur elle partage vos orientations politiques ; elle a même aggravé le texte en exonérant les industriels du médicament et en repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans.

son travail. Après une semaine d'échanges passionnants sur les finances de notre système de sécurité sociale, il nous revient de conclure l'examen de ce nouveau PLFSS. C'est avec un sentiment partagé que le groupe Union Centriste aborde le vote de ce projet de loi. loi. Nous reconnaissons plusieurs avancées : la gratuité de la contraception féminine jusqu'à vingt-cinq ans, l'instauration d'un tarif plancher pour la rémunération des aides à domicile et l'élargissement du champ des personnels concernés par le Ségur

Notre groupe salue la décision de la rapporteure générale de supprimer la trajectoire financière pluriannuelle de la sécurité sociale présentée par le Gouvernement. Monsieur le ministre, vous prévoyez de très lourds déficits au moins jusqu'en 2025, sans aucune stratégie de retour à l'équilibre. Cela n'est pas acceptable ! La La dette publique inquiète. Elle inquiète nos concitoyens les plus âgés comme les plus jeunes, lesquels se demandent s'ils toucheront un jour une retraite et s'ils pourront profiter des mêmes services publics que leurs parents et leurs grands-parents.

visuels et la prescription de corrections optiques. L'ajout de l'avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie pour étudier les textes d'application nous semble être une mesure de bon sens.

Bien trop de professionnels ne sont pas concernés par les augmentations de salaire prévues par le Ségur de la santé- nous les avons reçus, les uns et les autres, dans nos permanences. Ce n'est pas normal et c'est même, pour certains d'entre eux, profondément injuste.

sommes de fervents défenseurs du paritarisme et du dialogue social. Il est urgent de définir de nouvelles modalités de revalorisation salariale équitables dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. La quatrième mesure qui nous tient particulièrement à coeur est l'accès aux soins dans les milieux ruraux, et notamment la réduction de la fracture avec les milieux urbains. Une étude publiée par l'Association des maires ruraux de France (AMRF) dresse, chiffres de l'Insee à l'appui, un constat alarmant : les Français vivant dans les départements

à combler, année après année, les déficits de la sécurité sociale ! Très bien ! . Je regrette ce manque d'ambition en matière de politique familiale, à l'exception de la systématisation de l'intermédiation des pensions alimentaires. Le taux de natalité dans notre pays est en chute constante depuis près de dix ans. Nos politiques, initialement universalistes, ont été détricotées sous couvert d'une fausse justice sociale. Une proposition de loi pour revenir sur l'universalité de nos politiques sociales sonne donc comme une urgence- je m'engage à la déposer.

Il y a un an, nous constations tous avec effroi les conséquences désastreuses de la pandémie sur les comptes sociaux, qui approchaient jusque-là l'équilibre.

et des retraites. Ce PLFSS est le dernier du quinquennat. Il porte en lui quelques marqueurs positifs de la politique de santé promue par le Gouvernement, tels que les revalorisations salariales des personnels des secteurs sanitaire et médico-social ou l'innovation et la sécurité de l'approvisionnement en médicaments. Que peut-on attendre du dernier PLFSS d'un quinquennat ? Pas de grandes annonces. Il est censé clore l'exercice, boucler la boucle. Il apparaît ainsi logique de renvoyer au prochain gouvernement le soin d'envisager les mesures fortes, les réformes d'ampleur, les projets de long terme. Je pense, bien évidemment, à la grande loi sur l'autonomie, nécessaire et urgente, que l'on attendait. Ce PLFSS comporte toutefois quelques mesures intéressantes, permises

et la production en Europe de molécules stratégiques. Si nous regrettons tous que la loi sur le grand âge n'ait pu voir le jour, nous trouvons dans ce PLFSS quelques mesures satisfaisantes comme les recrutements dans les Ehpad, la revalorisation de l'allocation journalière du proche aidant ou l'instauration d'un tarif plancher à 22 euros par heure de prestations d'aide à domicile pour les personnes handicapées et en perte d'autonomie. Ce secteur avait, lui aussi, un grand besoin de revalorisation. Par ailleurs, l'assurance maladie prendra désormais en charge la contraception pour toutes les femmes de moins de vingt-six ans. Nous sommes toutefois nombreux à regretter que cette prise en charge ne s'étende pas aux jeunes hommes : la contraception masculine fait l'objet de nouvelles méthodes efficaces qu'il serait bon de promouvoir, pour un juste partage de cette responsabilité entre les hommes et les femmes. Enfin, l'accès direct à certaines professions paramédicales a fait couler beaucoup d'encre. Je suis personnellement favorable aux mesures qui permettent de faire évoluer leurs missions et de libérer du temps médical. La médecine de ville est en crise, tout autant que l'hôpital. Malgré l'augmentation du nous avons devant nous une situation particulièrement inquiétante, et je pèse mes mots. Le manque de médecins se confirme et s'aggrave. Nous devons donc accepter ces mesures qui permettent d'accéder directement à un kinésithérapeute ou à un orthophoniste, lesquels sont souvent plus à même de définir le plan de soins dans leur domaine de compétences ou encore d'accéder à la prescription d'un infirmier en pratique avancée ou d'un orthoptiste pour des lunettes. Les précisions apportées par le Sénat me semblent aller dans le bon sens, sans remettre en cause ces avancées. À l'inverse, je suis opposée, comme la majorité de mon groupe, à toute forme de coercition, car celle-ci n'a jamais fait la preuve de son efficacité. Nous lui préférons la poursuite de la nécessaire transformation de l'organisation des soins, que l'option des zones franches médicales, adoptée lors des débats la semaine dernière, qui crée une exonération de cotisations sociales pour les généralistes et spécialistes s'installant dans des zones sous-dotées. Cette solution pourrait notamment être reprise dans les territoires frontaliers, où les soignants sont littéralement « aspirés » par les pays voisins qui rémunèrent davantage et offrent des conditions de travail bien meilleures. C'est particulièrement le cas au Luxembourg, où les soignants sont payés jusqu'à trois fois plus de l'autre côté de la frontière. Si la crise est encore trop présente pour lancer les réformes structurelles, nous avons appuyé la position de la commission s'agissant de l'équilibre général des comptes de la sécurité sociale. Il n'est pas normal que la gestion d'une pandémie par l'État plombe aussi durablement et durement nos comptes sociaux. Il en est de même pour la reprise de la dette hospitalière : elle devrait être portée par le budget général de l'État et non par la sécurité sociale. Il manque une réflexion de fond et des propositions sur le retour à l'équilibre financier. Nous nous en étions rapprochés avant la crise sanitaire. Mais, d'une part, c'était le résultat de trop longues années de baisse des budgets des hôpitaux, de manque d'investissement, de retard dans les recrutements, les conditions de travail et la rémunération. Or, comme l'a souligné M. le ministre, « nous ne reviendrons pas aux méthodes du passé ». Nous ne le pouvons pas ! Néanmoins, il est nécessaire de renforcer le travail d'efficience sur les dépenses de santé pour faire que chaque euro dépensé le soit pour de bonnes raisons. D'autre part, il faudra diversifier les sources de financement, car d'autres crises sanitaires et écologiques pourraient survenir, et mettre définitivement en péril notre système de santé. Nous ne pouvons pas vivre éternellement à crédit et nous contenter d'un déficit chronique, estimé encore à 15 milliards d'euros en 2025. La refonte de notre système de santé doit être au coeur des préoccupations de cette campagne électorale. La crise nous a rappelé l'importance de préserver un système de soins performant. La santé est revenue sur le devant de la scène depuis bientôt deux ans. Et, puisque tout est désormais politique à l'approche de l'élection présidentielle, j'en appelle aux candidats pour qu'ils s'engagent à consolider notre modèle en misant notamment sur nos équipes soignantes,

Bien que la plupart d'entre nous considèrent comme nécessaire une réforme des retraites, nous n'avons pas soutenu l'introduction de mesures structurelles dans ce PLFSS. Comme pour la question de l'autonomie,

Monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai très bref. Je veux tout d'abord saluer l'ambiance de travail, à la fois précise,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que la COP26 vient de s'achever, la France est confrontée à une crise énergétique inédite, qui risque de l'éloigner de l'objectif de neutralité carbone issu de l'Accord de Paris de 2015 et de la loi du 8 novembre 2019 Il s'agit d'une triple crise : du prix des énergies, du système énergétique, mais aussi de la décision politique. La flambée du prix des énergies est sans précédent. Entre 2020 et 2021, les prix de marché ont été multipliés par deux pour le gaz, par trois pour le pétrole et par neuf pour l'électricité. Cette hausse s'est répercutée sur les tarifs réglementés, avec une augmentation de 12 % pour le gaz, en octobre, et de 4 % pour l'électricité, en février. Or cette flambée était prévisible : dès juin 2020,

Cette flambée pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, car l'énergie représente 10 % de leur budget. Selon le médiateur national de l'énergie, 95 % des ménages constatent une hausse, 60 % restreignent leur chauffage et 25 % diffèrent leurs paiements. cette baisse du pouvoir d'achat pourrait se muer en hausse de la précarité énergétique, laquelle affecte d'ores et déjà 3,5 millions de ménages. Cette flambée pèse aussi sur les coûts de production des entreprises, mettant en danger leur rentabilité économique et leur viabilité financière. C'est le cas des 400 entreprises énergo-intensives. Parce qu'elles consomment la moitié de l'énergie du secteur de l'industrie, le surcoût pourrait s'élever pour elles à plus de 1 milliard d'euros À terme, cette flambée désorganise le marché de l'énergie. Les litiges se multiplient déjà entre consommateurs et fournisseurs, et l'activité du médiateur a crû de 15 % en six mois. Certains fournisseurs font d'ailleurs défaut. Or les fournisseurs de secours, qui auraient dû être désignés depuis bientôt deux ans, en application de la loi Énergie et climat, l'ont été la semaine dernière pour l'électricité ... Et leur désignation est encore attendue pour le gaz ! Outre cette flambée, notre système énergétique est Notre sécurité d'approvisionnement se dégrade. Réseau de transport d'électricité (RTE) a placé la France en situation de « vigilance particulière » sur la période 2021-2024.

Notre transition énergétique stagne. Les objectifs liés aux énergies renouvelables, fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, ne sont pas atteints. Selon RTE, l'écart est de 53 % pour le photovoltaïque, de 25 % pour l'éolien et de 1 % pour l'hydroélectricité. Les objectifs liés aux émissions de CO2, issus de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), ne le sont pas non plus. Pour le Haut Conseil pour le climat (HCC), le premier budget carbone a ainsi été dépassé de 62 millions de tonnes. Notre avenir énergétique se complexifie. Dans son étude intitulée , RTE s'est inquiété des deux défis auxquels la France sera confrontée l'électrification des usages, de 15 à 60 % supplémentaires, et le renouvellement du parc nucléaire, avec un « effet falaise » dès 2040 Dans ce contexte très dégradé, la politique énergétique du Gouvernement est marquée du sceau de l'indécision. En premier lieu, le « bouclier tarifaire » est tardif et limité. L'attribution de 100 euros le chèque énergie ou l'indemnité inflation est dérisoire, les prix à la pompe dépassant 1,50 euro par litre. Ces 100 euros sont l'équivalent d'un plein, et non une solution pérenne pour passer l'hiver ! Les tarifs réglementés, sur lesquels se focalisent les blocages ou compensations de prix, ne concernent que 7,5 % de la consommation nationale de gaz et 28 % de celle d'électricité. Les entreprises énergo-intensives ne bénéficient que d'une avance de 150 millions d'euros, une aide six fois inférieure aux besoins Enfin, les baisses de taxes sur la consommation d'énergie sont facultatives, activables par décret et transitoires, limitées à un an.

les réformes énergétiques sont embourbées. Le projet Hercule, la réforme de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, le règlement du contentieux sur les concessions hydroélectriques tous ces chantiers ont été suspendus, faute d'accord avec la Commission européenne. Le Gouvernement doit clarifier ses intentions ! Sur ce sujet, je veux dire solennellement

Si je prends acte de l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs, je vous le demande : pourquoi avoir attendu si longtemps ? Et pourquoi avoir fermé les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim en 2020 ? ? Je prends acte, aussi, de l'annonce de 500 millions d'euros consacrés aux petits réacteurs modulaires, mais elle est largement en deçà de la politique stratégique menée par les États-Unis ou le Royaume-Uni. Surtout, pourquoi avoir fermé le démonstrateur Astrid en 2019

Une politique énergétique, nucléaire, ne s'improvise pas ; elle s'anticipe. Et elle ne peut souffrir d'effets d'annonces, car le montant et la durée des investissements sont colossaux. Alors, passons des annonces aux décisions ! Nous attendons que le Gouvernement indique s'il compte relever la part de 50 % d'énergie nucléaire. Je regrette qu'il n'ait pas demandé à RTE de tester un scénario supérieur à cette proportion. Nous souhaitons que le Gouvernement fasse savoir s'il compte revenir sur la trajectoire de fermeture des réacteurs existants. Je rappelle que RTE, dans son scénario

que le Gouvernement reprenne l'effort de recherches en direction de la fermeture du cycle du combustible, et qu'il soutienne le très prometteur projet ITER (). Il faut lancer des plans de relance et d'investissement. Enfin, nous appelons le Gouvernement à veiller à l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte. Il serait incompréhensible que le gaz fossile y soit intégré et non le nucléaire,

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse de représenter aujourd'hui le Gouvernement pour aborder cet enjeu crucial de la souveraineté énergétique de la France. Barbara Pompili m'a chargée de la représenter, puisqu'elle est en ce moment même en déplacement aux côtés du Président de la République pour promouvoir la filière hydrogène. Pour faire évoluer notre mix énergétique et atteindre la neutralité carbone en 2050, le Gouvernement s'est fixé une ligne claire - j'ai même presque entendu dire qu'elle était « incontestable » dans le discours précédent Le levier essentiel pour renforcer notre souveraineté énergétique consiste à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Ces énergies fossiles importées représentent près des deux tiers de notre consommation énergétique, 63 % pour être exacte,

présentent plusieurs options, mais une constante apparaît dans tous les scénarios : la neutralité carbone en 2050 suppose d'ici là une sortie des énergies fossiles. Si cet horizon peut paraître lointain, c'est dès aujourd'hui que nous devons préparer l'avenir. préparer l'avenir. La stratégie du Gouvernement est claire. Elle repose sur un triptyque : efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, relance du nucléaire. nucléaire. Pour sortir des énergies fossiles, le premier pilier de notre action consiste en la sobriété énergétique et en la réduction globale des consommations d'énergie, en complément des mesures de soutien au pouvoir d'achat que nous avons mises en place avec l'augmentation du chèque énergie de 100 euros,

conformément à la stratégie nationale bas-carbone. Il s'agit d'un défi d'une ampleur considérable, mais nous sommes actuellement sur le bon chemin, notamment grâce aux politiques menées depuis 2017, qui commencent à porter leurs fruits.

Nous avons aussi mis en place un soutien à des projets d'efficience énergétique dans l'industrie. Toutefois, pour sortir des énergies fossiles, et parallèlement à la réduction de notre consommation totale d'énergie, il faudra électrifier divers usages dans la mobilité, le chauffage ou encore l'industrie.

L'électricité viendra ainsi remplacer les énergies fossiles importées, avec un effet positif sur notre indépendance énergétique comme sur nos émissions de gaz à effet de serre.

Pour relever ce défi, le deuxième pilier de l'action gouvernementale consiste à accélérer le développement des énergies renouvelables (EnR). Nous avons déjà progressé : aujourd'hui, 25 % de notre électricité est produite par des EnR, contre 21 % en 2018. Mais il sera nécessaire de doubler les capacités de production d'EnR d'ici à 2030, et de les accroître encore davantage d'ici à 2050. Nous devons donc accélérer le développement de toutes les énergies renouvelables dès aujourd'hui pour tenir nos objectifs de décarbonation, en particulier lors des quinze prochaines années, au cours desquelles la capacité de production nucléaire va décroître avec l'arrivée en fin de vie d'une partie du parc, avant la mise en service de nouvelles centrales. Sur l'éolien terrestre, il nous faudra atteindre en 2050 entre deux et quatre fois la capacité actuellement installée, pour atteindre alors plus ou moins le niveau d'équipement actuel de l'Allemagne. Nous devons également développer massivement l'éolien en mer, avec pour objectif d'avoir mis en service entre 2 000 et 4 000 éoliennes offshore à l'horizon de 2050. Nous déploierons également le photovoltaïque, en visant une multiplication entre sept et douze des capacités installées d'ici à 2050, ce qui mobilisera plusieurs dizaines de milliers d'hectares de toitures et de sols, dans le respect de nos objectifs de lutte contre l'artificialisation Au-delà du système électrique, le biogaz sera aussi une énergie importante, en se substituant progressivement au gaz naturel pour les usages résiduels. L'objectif est que le biogaz représente au moins 10 % du gaz consommé en 2030, contre 1 % aujourd'hui. En somme, l'ensemble des énergies renouvelables jouera un rôle essentiel pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais notre souveraineté énergétique passe également par la constitution de filières industrielles compétitives en France. Avec le plan France Relance, nous mobilisons 7 milliards d'euros pour développer l'hydrogène décarboné. Pour aller plus loin encore, le plan d'investissement France 2030 prévoit des soutiens complémentaires envers la filière hydrogène, mais aussi les EnR et l'intégration des systèmes énergétiques. Le nucléaire est le troisième pilier de notre politique de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, il est largement majoritaire dans notre mix électrique. À l'horizon de 2050, il en constituera encore un socle important en complément des énergies renouvelables. RTE confirme dans son rapport que la relance des capacités de production nucléaire permettra aux Français de disposer à l'horizon de 2050 d'une électricité compétitive. Le Président de la République a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, en invitant la filière industrielle à s'y préparer. L'objectif est de permettre, à partir de 2035, la poursuite de l'électrification des usages et le remplacement d'une partie des réacteurs existants qui arriveront en fin de vie. Si la part du nucléaire dans le mix électrique décroîtra mécaniquement au fil des fermetures des réacteurs, la mise en service de nouveaux réacteurs, débutant dans une quinzaine d'années, permettra de conserver un socle significatif de nucléaire de manière à optimiser notre mix. Mesdames, messieurs les sénateurs, voilà la ligne du Gouvernement. Mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles et renouveler nos capacités de production électrique est un réel défi, comme nous n'en avons pas connu depuis un demi-siècle. Mais c'est aussi une opportunité historique pour renforcer l'indépendance énergétique de notre pays et la résilience de notre économie. Je sais qu'ensemble, nous saurons la saisir. Nous allons

nous partageons tous et toutes, dans cet hémicycle, l'idée que la reconquête d'une souveraineté énergétique constitue un enjeu majeur pour notre pays. La question à laquelle nous devons répondre à travers ce débat est celle des leviers pour la rendre effective. La privatisation des acteurs du secteur de l'électricité et le démantèlement des opérateurs publics historiques ont conduit à une perte de contrôle de l'État sur la production et la distribution de l'énergie. Les conséquences pour les consommateurs ne sont pas celles qui avaient été promises : même sans compter les dernières envolées des prix, les tarifs de l'électricité ont augmenté de 60 % depuis l'ouverture du marché en 2007. L'État, démuni face à la volatilité structurelle de ce marché, en est réduit à devoir sortir son carnet de chèques à chacun de ces dérapages. Pour certaines énergies, comme le gaz, nous sommes même devenus dépendants de pays étrangers.

De même, ce service public serait le mieux placé pour relever l'indispensable défi du développement des énergies renouvelables. Le développement anarchique de projets conduits par des acteurs privés sans tenir compte des intérêts des territoires concernés suscite une résistance grandissante chez nos concitoyens. Deux exemples de projets d'installation d'éoliennes dans mon département de la Loire me semblent très parlants. D'un côté, un projet à proximité des communes de Cherier, La Tuilière et Saint-Just-en-Chevalet, provoque une véritable résistance des élus locaux des élus locaux et de la population. C'est un groupe énergétique étranger qui le porte, dans un total déni de démocratie. De l'autre côté, le projet des « Ailes de Taillard », sur les communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue, porté dans une démarche participative par la communauté de communes, une association citoyenne et un acteur industriel, a permis d'obtenir une vraie adhésion des riverains. C'est bien ce second type de modèle qu'il faut suivre pour donner une nécessaire acceptabilité à cette énergie : un projet pensé avec les citoyens et les élus, dont le territoire cher collègue. ... quel que soit le nom que vous voudrez lui donner, envisagez-vous, madame la ministre, d'aller vers ce service public de l'énergie, outil majeur pour une reconquête de la souveraineté énergétique de notre pays

Certaines sont d'ailleurs dans la droite ligne de la loi Climat et résilience, lors de l'examen de laquelle a été votée la mise en place de commissions régionales de l'énergie qui permettront

5,8 millions de ménages vont bénéficier le mois prochain d'un chèque énergie exceptionnel de 100 euros, et c'est une bonne nouvelle. Entre partisans du nucléaire et défenseurs des énergies renouvelables, la politique énergétique du Gouvernement est équilibrée. Celle-ci repose, d'une part, sur le développement des énergies renouvelables et, d'autre part, sur le rôle essentiel accordé au nucléaire. Cette position équilibrée a été rappelée la semaine dernière par le Président de la République.

Lors de la présentation du plan France 2030, un investissement de 1 milliard d'euros a été annoncé pour le développement de technologies de rupture dans le domaine du nucléaire. Cela passe par le développement de réacteurs de petite taille,

que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinente, je voudrais savoir, madame la ministre, quelle place peuvent occuper les SMR dans les années à venir pour favoriser notre souveraineté énergétique. Comment ces projets vont-ils se coordonner

Ces atouts pourraient permettre aux SMR de venir compléter une offre nucléaire de grande puissance. Ils sont aussi susceptibles de répondre aux besoins de sites isolés ou de zones dans lesquelles le développement du réseau électrique est insuffisant.

La relance à court terme d'un nouveau programme nucléaire en France reposera sur des technologies éprouvées telles que l'EPR. Le SMR français pourra compléter dans un second temps l'offre nucléaire du mix énergétique, dans le cadre d'un déploiement industriel à l'horizon 2040.

Elle nous permet d'obtenir une électricité décarbonée et nous assure une production stable dont nous conservons le contrôle. Le contexte géopolitique actuel nous rappelle que l'indépendance énergétique est un vrai levier de souveraineté et même d'indépendance politique.

Dès son adoption, je faisais partie de ceux qui doutaient de son réalisme et de son équilibre sur le long terme. Force est de constater que notre politique énergétique doit souvent faire face à des injonctions contradictoires. La fermeture de la centrale de Fessenheim, guidée plus par des considérations politiques que par des réalités techniques ou de sûreté, en est le parfait exemple. Bien sûr ! Elle fait peser le risque de tensions sur notre approvisionnement et nous contraint à repousser par là même la fermeture des dernières centrales à charbon. En effet, RTE vient de publier des scénarios à l'horizon de 2050 qui font apparaître qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, même avec un développement très ambitieux et nécessaire des énergies renouvelables dans le cadre des usages électriques.

Ne mérite-t-elle pas aussi un ministère dédié, afin de porter une véritable politique énergétique cohérente et de long terme ?

de l'usage des énergies fossiles. C'est dans ce cadre qu'a été pilotée la fermeture des quatre dernières centrales à charbon. Deux sont déjà très engagées, au Havre et à Saint-Avold.

La loi relative à l'énergie et au climat promulguée en novembre 2019 prévoit qu'une loi de programmation de politique énergétique et climatique sera adoptée d'ici à la mi-2023, puis que la PPE sera adaptée un an plus tard, soit à la mi-2024. La prochaine PPE couvrira les périodes 2024-2033. Le Parlement sera donc étroitement associé aux choix énergétiques à l'avenir, en application, donc, de la loi Énergie et climat. Afin d'alimenter les réflexions, le Gouvernement a lancé le 2 novembre dernier une concertation ouverte à tous sur internet autour de douze grands thèmes de la stratégie française sur l'énergie et sur le climat. Depuis le début du mois de novembre, les premiers groupes de travail technique avec les parties prenantes ont démarré. Ils se poursuivront jusqu'à l'automne 2022. À l'issue du débat parlementaire sur la loi de programmation, la PPE fera l'objet au deuxième semestre 2023 d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant et de la Commission nationale du débat public. Comme vous le voyez, le Parlement sera désormais totalement associé aux grands choix énergétiques français.

collègue ministre de l'économie, qui propose de réformer le marché européen de l'énergie. C'est une excellente idée, mais il faudrait être un petit peu plus précis et plus clair sur les ambitions du Gouvernement, à condition naturellement d'être certain que le ministre parle bien au nom de celui-ci ... En matière de souveraineté énergétique

en faisant appel à chaque instant au moyen de production le moins cher à l'échelle de la plaque européenne, au bénéfice de l'ensemble des consommateurs. Comme les marchés sont interconnectés à l'échelle européenne, c'est donc le prix du dernier moyen de production appelé dans l'ensemble de l'espace qui établit le prix du marché. En ce moment, il s'agit en général d'une centrale au gaz, ce qui lie le prix de marché de l'électricité au prix du gaz. Cette situation persistera probablement tant que les moyens de pointe fossiles seront nécessaires pour assurer l'équilibrage du système. La persistance de prix élevés sur ces marchés est préoccupante. C'est la raison pour laquelle la France plaide pour une évolution de l'articulation entre l'amont et l'aval du marché européen de l'électricité, pour que le prix payé par le consommateur reflète les coûts de production du système électrique et du mix national, et non le prix marginal fossile. La France estime que cette démarche est tout à fait compatible avec le fonctionnement du marché européen de gros. L'ensemble du Gouvernement - je vous rassure sur ce point - est très mobilisé pour faire avancer ce sujet crucial

prix payé par les consommateurs et le coût de production de la composante bas-carbone du mix électrique national. Nous souhaitons également introduire dans la directive européenne le droit pour les consommateurs d'avoir accès à des contrats de fourniture d'électricité

la taxonomie, à condition que vous obteniez en effet des résultats. Je vous rappelle que le système du coût marginal calculé sur la dernière centrale à charbon ou à lignite allemande est simplement absurde. S'il y a des pays européens qui refusent l'énergie moderne et décarbonée, c'est leur problème, et ils n'ont pas à nous le faire payer

qui soient renouvelables et compétitifs, qui contribuent à notre indépendance énergétique et qui renforcent la résilience de notre système électrique. La faisabilité technique d'un mix électrique électrique décarboné, sans nouveau nucléaire, 100 % renouvelable, d'ici à 2050, est possible ! Si certains aiment accuser l'éolien de tous les maux, il est pourtant l'une des clés majeures de la transition.

d'une filière qui crée de l'activité économique et de l'emploi sur tout le territoire, du sous-traitant au développeur-exploitant, en passant par les bureaux d'études, l'ingénierie ou les constructeurs de turbines. Aujourd'hui, en France, le tissu industriel éolien regroupe plus de 900 entreprises et près de 23 000 emplois. Les perspectives et les opportunités des prochaines années sont immenses. Concernant l'éolien en mer, le premier parc offshore situé à Saint-Nazaire va être inauguré dans quelques mois, vingt ans après ceux des Anglais, des Belges ou des Danois Danois ! Notre pays est pourtant idéalement configuré pour son développement, puisqu'il possède la deuxième surface maritime mondiale, avec quelque 11 millions de kilomètres carrés de zone maritime. Globalement, l'éolien montre un retard préoccupant sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Sans même aller jusqu'à un scénario d'énergies 100 % renouvelables, les objectifs de la PPE nous somment d'atteindre en capacité installée le double de la situation actuelle. Dans les six prochaines années, nous devons passer de 17,8 gigawatts en 2021 à 34,1 gigawatts en 2028. L'État doit être davantage proactif dans l'accompagnement de cette énergie nouvelle. Comment, madame la ministre, la puissance publique compte-t-elle agir pour rattraper ce retard et favoriser un développement harmonieux dans les territoires ? La parole est à Mme la ministre

il nous faudra développer de façon très volontariste toutes les énergies renouvelables, y compris l'éolien terrestre et l'éolien en mer. L'éolien terrestre contribue déjà à la lutte contre le réchauffement climatique. RTE a calculé qu'en 2019, les parcs photovoltaïque et éolien français ont permis d'éviter l'émission de 22 millions de tonnes de CO2 en se substituant à des moyens fossiles. L'éolien contribue aussi à notre sécurité d'approvisionnement. En 2020, l'éolien terrestre a représenté 8 % de notre production électrique nationale, ce qui en fait la troisième source derrière le nucléaire puis l'hydroélectricité, et devant les centrales à gaz. Enfin, il crée des emplois sur notre territoire. La filière éolienne représente plus de 22 000 emplois directs et indirects à la fin de 2020. Le Gouvernement souhaite donc poursuivre le développement de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer pour atteindre les objectifs ambitieux de la PPE. À cette fin, pour le terrestre, nous avons mis en place cet été un nouveau dispositif d'appels d'offres pour la période 2021-2026, qui permettra de lancer au moins 25 gigawatts de nouveaux projets terrestres photovoltaïques et de petite hydroélectricité durant les cinq années à venir. Nous travaillons bien sûr à maintenir l'acceptabilité des énergies renouvelables. La ministre de la transition écologique a ainsi annoncé, au début du mois, dix mesures pour garantir un développement responsable de l'éolien terrestre, dont la mise en place d'un médiateur de l'éolien, des contrôles systématiques du bruit, des expérimentations pour réduire les nuisances liées au balisage, ou la création d'un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel alimenté par les développeurs éoliens.

en continuant de vendre nos fleurons industriels énergétiques et en voulant démembrer l'entreprise historique, EDF ? La parole

développer massivement les énergies renouvelables, les capacités de stockage ainsi que les réseaux intelligents. La priorité du Gouvernement est qu'EDF dispose de capacités accrues d'investissement pour qu'elle puisse participer pleinement à la transition énergétique dans ses différentes composantes, tout en restant une entreprise intégrée et publique. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de l'État, consistant à sécuriser le maintien des installations nécessaires au succès de nos ambitions climatiques afin de corriger, je l'indiquais, les imperfections du marché de l'électricité.

pour investir, notamment dans la filière nucléaire et dans la transition énergétique ! Il faut conclure. Bref, vous faites exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour conquérir la souveraineté énergétique française, c'est-à-dire sortir le secteur de l'énergie des mains

La poursuite de l'essor des énergies renouvelables est une première partie de la réponse, comme le démontre le rapport de RTE publié le 25 octobre dernier, mais la relance du nucléaire est l'autre pendant de la réponse. Alors que, depuis les années 1970, l'énergie nucléaire a contribué à éviter, à l'échelle mondiale, l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de 63 gigatonnes de CO2, de CO2, il serait impensable de ne pas s'appuyer sur cette énergie pour décarboner et électrifier notre économie et il serait plus que regrettable qu'elle ne figure pas dans la taxonomie européenne. les dernières annonces présidentielles vont dans le bon sens et permettent de replacer l'atome au coeur de la transition énergétique, mais nous ne pouvons que déplorer le temps perdu dans ce secteur pourtant crucial.

cet engagement nous oblige. Dans ce contexte, je m'interroge sur le projet de renouvellement d'un tiers de nos contrats de concessions hydroélectriques en 2023 et de possibles ouvertures de ces ouvrages à la concurrence, à la découpe. Compte tenu des besoins croissants, la tentation est en effet grande de privatiser ces concessions et d'accélérer à tout va la production hydroélectrique, sans respecter les multiples usages partagés : le loisir, l'approvisionnement local et les usages agricoles. Les acteurs de l'hydroélectricité s'inquiètent légitimement du changement de gouvernance, radical, technocratique et totalement libéralisé, qui pourrait se profiler. Madame la ministre, à quelques jours de la présidence française de l'Union européenne et, il faut le rappeler, ans après la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), quelles initiatives européennes comptez-vous prendre pour assurer la protection de notre modèle national de production hydroélectrique, qui fait la fierté de notre pays ? La parole est à Mme la ministre

tant que ministre chargée du logement, je mène avec les associations un travail sur la lutte contre la précarité énergétique, notamment en faisant en sorte que les ménages les plus modestes puissent avoir accès à des bouquets de travaux qui leur permettent de rénover leur logement et en incitant les propriétaires bailleurs à rénover les passoires thermiques. En effet, en général,

le droit français, les concessions hydroélectriques échues doivent être renouvelées par mise en concurrence. Or plusieurs concessions sont arrivées à échéance entre la fin de 2011 et aujourd'hui, sans que la procédure concurrentielle ait été engagée, les gouvernements successifs s'étant donné le temps de préparer la mise en concurrence avec l'ensemble des acteurs.

Cette situation nuit aux investissements dans le secteur, elle est source d'incertitude pour les entreprises, les salariés et les collectivités. C'est pourquoi le Gouvernement a engagé des discussions avec la Commission européenne pour trouver une solution. Dans le cadre des réflexions menées autour de la réorganisation du groupe EDF, le Gouvernement explore également la voie consistant à attribuer sans mise en concurrence les concessions à une structure publique dédiée, contrôlée par l'État ; c'est le régime de la quasi-régie, qui s'accompagne d'exigences fortes faisant l'objet d'échanges avec la Commission. Aucun accord n'a encore été trouvé,

qui se répercutent sur les coûts de production. Bien que, en France, cela ne représente que 6 % de l'électricité produite, la libéralisation du marché européen de l'énergie affecte les factures des particuliers et des entreprises, et remet en cause notre indépendance énergétique. Nous dépendons en effet de l'extérieur pour nous approvisionner en énergies fossiles et en uranium, dont nous importons la totalité de nos besoins, soit 9 000 tonnes par an. Pour gagner en indépendance énergétique et géopolitique, faire face aux fluctuations de prix ainsi qu'au risque de pénurie et de énergétique, nous devrions stocker notre propre électricité. Or, à l'heure actuelle, l'énergie produite par les barrages hydroélectriques est la seule stockable ; elle est également non émettrice de CO2, 100 % renouvelable et très compétitive, puisque les barrages produisent une électricité à 30 euros par kilowattheure. Miser sur cette énergie réduirait donc notre dépendance et permettrait d'avoir une stratégie affinée en matière de pilotage du système électrique. Elle soutiendrait notamment les entreprises électro-intensives, qui doivent bénéficier d'une énergie peu coûteuse.

l'Union des industries utilisatrices d'énergie (Uniden) prévoit une hausse d'un tiers de la facture d'électricité des industries françaises. Du reste, outre l'industrie, tous les secteurs économiques sont touchés, d'une façon ou d'une autre. À cette hausse, déjà susceptible de créer un déficit concurrentiel vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, s'ajoute une augmentation du prix des matières premières. Or préserver la souveraineté énergétique de la France n'a de sens que si l'on préserve aussi la compétitivité de nos entreprises, qui attendent du Gouvernement une vision à long terme,

Il est donc urgent de mettre en place une politique énergétique qui sécurise les approvisionnements, les tarifs, mais également les finances publiques. Aussi, madame la ministre, comment allez-vous préserver notre souveraineté énergétique, gage de la compétitivité de l'ensemble des entreprises françaises ? La parole

inédite depuis la création du marché européen de l'énergie, avec une augmentation des prix sans précédent qui s'applique à tous les pays d'Europe et qui est principalement liée à une très forte hausse des prix du gaz naturel.

ce bouclier tarifaire sur l'électricité bénéficiera aussi aux entreprises, dans la limite d'un taux minimal de 0,50 euro par mégawattheure prévu par le droit communautaire. Pour les entreprises les plus électro-intensives,

Cette augmentation permettra de renforcer en cours d'année la trésorerie des entreprises, alors que ces dernières connaissent actuellement une forte hausse de leur facture énergétique, notamment d'électricité, quand elles s'approvisionnent sur le marché. En outre, les entreprises bénéficient d'un cadre réglementaire plus protecteur que leurs principaux concurrents européens, grâce à l'Arenh, une spécificité française bénéficiant à tous les consommateurs et permettant aux entreprises d'être protégées des fluctuations de prix de marché pour une part importante de leur approvisionnement électrique.

Les entreprises françaises ont quasiment un seul avantage concurrentiel : le prix de l'énergie. C'est pour cette raison qu'il faut être d'une grande vigilance. Je vous remercie donc des quelques annonces que vous faites, mais il faut aller très vite, afin d'éviter de perdre, encore une fois, notre place sur les marchés internationaux.

la COP26, qui vient de s'achever, nous rappelle l'urgence qu'il y a à accentuer nos efforts en faveur d'un mix énergétique décarboné visant à limiter les dégâts du dérèglement climatique. Le récent rapport de RTE fournit deux axes de réponse : investir massivement dans les EnR et, en parallèle, au moins maintenir, si ce n'est accroître, notre production d'électricité nucléaire. À ce titre, je tiens à saluer les choix récents du Gouvernement en faveur de cette filière, avec le plan de relance France 2030, visant à financer de petits réacteurs modulaires, que l'annonce, par le Président de la République, de la construction de nouveaux réacteurs EPR. Ce n'est pas trop tôt ! En effet, alors que de nombreuses centrales vont être mises en maintenance pour prolonger leur fonctionnement, l'intermittence des EnR nous place à la merci des productions d'énergie étrangères, qui ne sont pas toujours aussi vertueuses que nous du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour éviter ce scénario qu'il est nécessaire d'intensifier le développement des EnR, mais également de relancer immédiatement le nucléaire, afin de conserver notre souveraineté énergétique. Il sera alors particulièrement important de dialoguer avec les élus locaux, car les territoires, notamment ruraux, seront les premiers affectés par les aménagements nécessaires pour atteindre cet objectif. Il serait notamment

que la question sera posée, une fois que nous aurons précisé l'ambition du Gouvernement et du Président de la République. La Commission nationale du débat public enclenchera alors le débat public nécessaire et légitime sur la suite du développement du nucléaire en France. Côté énergies

les collectivités locales, lesquelles jouent, effectivement, un rôle important. À cet égard, Mme la ministre de la transition écologique a demandé aux préfets de région, en mai dernier, d'établir, en concertation avec les collectivités et toutes les parties prenantes, une cartographie des zones favorables au développement de l'éolien. Les premiers résultats seront disponibles à la fin de cette année et les cartographies seront finalisées d'ici à la mi-2022. La loi Climat et résilience accentue cette planification, en prévoyant une déclinaison régionale des objectifs, en matière d'EnR, de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette déclinaison sera établie en lien avec les régions et en consultant les nouveaux comités régionaux de l'énergie, qui regroupent notamment les collectivités et les principaux acteurs concernés. Ces dispositions permettront d'établir une planification au plus près des territoires

par notre capacité à respecter concrètement le mix énergétique global et la trajectoire de la PPE dans le temps. L'augmentation, probablement très importante, des usages domestiques et industriels de l'électricité pose donc la question de notre capacité nationale à disposer, en temps voulu, de tous les modes de production prévus. Cela vaut pour le nucléaire tout autant que pour les énergies renouvelables. Les problèmes que rencontrent aujourd'hui nombre de territoires pour développer des projets photovoltaïques ou de méthanisation,

Or on constate aujourd'hui que, dans nombre de territoires, le pilotage et l'organisation des parties prenantes sont inexistants ou insuffisants pour mener à bien les dossiers présentés.

rationaliser les processus d'autorisation des projets et, en définitive, être au rendez-vous, en temps voulu, des objectifs départementaux, régionaux et nationaux

C'est l'objet de la feuille de route que Mme la ministre Barbara Pompili a présentée récemment, qui comportait dix mesures pour l'éolien, à commencer par la demande expresse faite aux préfets d'être extrêmement vigilants à la cohérence territoriale et à l'acceptabilité des projets passant par le guichet préfectoral.

Un réseau de conseillers sur le photovoltaïque et l'éolien sera également mis en place, afin de soutenir les collectivités dans le développement de leurs projets. En parallèle de ces actions, pour améliorer la concertation et l'implication des collectivités et pour donner aux préfets un rôle renouvelé en matière d'énergies renouvelables, un arrêté de 2020 renforce les exigences sur le recyclage des éoliennes, qui est aussi un sujet important. Cet arrêté rend ainsi obligatoire l'excavation complète des fondations et impose de travailler sur les nuisances lumineuses. Toutes ces mesures techniques, en associant mieux les élus sous l'égide du préfet, devraient permettre d'atteindre les objectifs ambitieux de la PPE en matière d'énergies renouvelables.

les critères pour optimiser le positionnement des unités sur le réseau de raccordement ? Quelles seront les recommandations pour le cadre de pilotage collectif départemental : société d'économie mixte, coopérative ou autre ? Comment

Je vous remercie, voilà un an, l'exécutif annonçait son plan Hydrogène : plus de 7 milliards d'euros pour soutenir cette filière, qui permet de décarboner l'industrie et les transports. Cet engagement était attendu, tant il permettra d'accélérer notre transition écologique tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des importations d'hydrocarbures. Passé l'effet d'annonce, il a toutefois fallu attendre la semaine dernière pour entendre le Président de la République déclarer le retour en grâce de l'énergie nucléaire. Nous étions nombreux à juger cette attente incompréhensible : plaider en faveur de l'hydrogène bas-carbone, c'est nécessairement avoir recours à des quantités massives d'électricité. Si cette conversion récente du chef de l'État constitue en soi une bonne nouvelle, le flou qui l'entoure doit rapidement être levé. Je m'associe pleinement à la demande formulée par nos collègues de la commission des affaires économiques, qui exigent de la clarté, en particulier sur les arrêts des réacteurs existants et sur la construction d'EPR ou de SMR.

L'argent ne suffira pas au développement rapide d'une filière hydrogène compétitive à l'international si nos partenaires européens ne considèrent pas le nucléaire comme un allié indiscutable de la transition écologique. Lui seul offre, à l'heure actuelle, une capacité de production d'hydrogène suffisante pour répondre à l'enjeu écologique, technologique et économique. Évitons, comme pour la production des batteries, de perdre la guerre sans mener la bataille. Madame la ministre, comment le Gouvernement compte-t-il s'y prendre pour convaincre ses partenaires européens et assurer, dans les plus brefs délais, cette indépendance technologique qui manque tant à la France ? La parole est à Mme la ministre

La stratégie française repose sur une production nationale d'hydrogène à partir de notre mix électrique décarboné, composé de nucléaire et d'énergies renouvelables, ce qui doit nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'importation d'hydrocarbures. La France veut atteindre une capacité de 6,5 gigawatts d'électrolyseurs installés installés en 2030. Cet objectif ambitieux est cohérent avec la disponibilité d'électricité bas-carbone, d'origine tant nucléaire que renouvelable, que nous prévoyons dans le cadre de notre politique pluriannuelle de l'énergie. La disponibilité d'une électricité bas-carbone, au-delà de 2030, est un enjeu bien identifié. Dans son étude, RTE analyse plusieurs évolutions possibles du marché de l'hydrogène décarboné et les conséquences sur les besoins en électricité. Ces études seront prises en compte avec le plus grand sérieux pour élaborer la prochaine PPE, après l'adoption de la loi qui vous sera soumise en 2023. L'une des priorités de la stratégie française pour l'hydrogène décarboné réside dans le soutien à la recherche, à l'innovation et au développement de compétences. À ce titre, la question de l'augmentation du rendement du processus d'électrolyse

Premier pays exportateur d'électricité d'Europe, la France fournit 30 % de l'électricité de l'Union européenne et permet de réduire d'autant la dépendance aux énergies fossiles. Ces dernières, comme le charbon, le fioul ou le gaz, voient leur demande s'accroître et leur prix augmenter. Les Français sont alors mécaniquement confrontés à une hausse généralisée du prix de l'énergie. Afin d'anticiper les besoins futurs en électricité, qui s'annoncent exponentiels, la France va devoir mettre en oeuvre de nouvelles capacités de production d'électricité.

et développer les microcentrales SMR, tout cela bien entendu dans le cadre d'un mix énergétique dans lequel le photovoltaïque et l'éolien ont toute leur place. Cependant, il est impératif que l'éolien, notamment offshore, ne soit pas implanté n'importe où, n'importe comment et à n'importe quel prix.

les observateurs peinent à identifier les réelles intentions de l'exécutif. En effet, l'annonce d'une relance de la construction de réacteurs est frappée d'un flou artistique particulièrement inadéquat dans ses considérations scientifiques et stratégiques. Dès lors, madame la ministre, nous comptons sur vous pour préciser un certain nombre de points. S'agirait-il des les fameux SMR évoqués voilà quelques semaines par Emmanuel Macron lui-même, ou bien d'EPR de deuxième génération, dont la puissance reste à préciser ? Ou s'agirait-il d'une orientation guidée par des éléments nouveaux dont le Président de la République ne disposait pas au début de son quinquennat ? Par ailleurs, puisque nous évoquons notre souveraineté énergétique, quelle est la position du Gouvernement

en 1991 et en 2006 ? Si le Président de la République vise effectivement un tel objectif, pouvez-vous nous expliquer la cohérence de l'abandon du programme de recherche Astrid sur les réacteurs à neutrons rapides, les réacteurs de quatrième génération, seuls à même de nous assurer une véritable indépendance grâce au stock considérable de plus plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri dont nous disposons sur notre territoire ? Madame la ministre, à défaut d'avoir été consulté dans ces processus de décision, le Parlement attend des réponses claires de votre part. La parole est à Mme la ministre déléguée.

de plusieurs décennies, sans pour autant avoir totalement disparu. En effet, les ressources en uranium naturelles sont aujourd'hui abondantes et disponibles à bas prix ; elles devraient le rester jusqu'à la seconde partie du XXI siècle.

Au regard de ces constats, et en raison de son coût élevé, le projet Astrid a été suspendu à la fin de 2019. Le Gouvernement a décidé de concentrer ses efforts sur le multirecyclage des réacteurs de troisième génération, dans la préfiguration d'un développement plus performant de nouveaux réacteurs, notamment en matière de gestion des déchets. Le plan France 2030 s'inscrit dans cette logique. Pour autant, la PPE prévoit le maintien d'un programme de recherche sur la quatrième génération, reposant sur un volet de simulation et sur un volet expérimental,

Madame la ministre, dans quelque domaine que ce soit, la souveraineté ne se construit pas sur le temps court, ni dans la précipitation, et encore moins à la faveur d'une campagne électorale. J'aurais aimé vous entendre reconnaître l'incongruité des

la souveraineté, notamment la souveraineté énergétique, est au coeur de tous les débats. La crise sanitaire a fait évoluer la plupart de nos paradigmes, et même les plus libéraux redécouvrent aujourd'hui les bienfaits de l'indépendance économique et industrielle. La hausse abrupte des coûts de l'énergie- gaz, pétrole, électricité -, qui était prévisible, nous oblige aussi à revoir nos politiques et à réhabiliter ce qui était vilipendé ces dernières années. Bien évidemment, je pense ici au nucléaire. nucléaire. Le Gouvernement a arrêté, en 2019, le projet de recherche sur les réacteurs de quatrième génération, décision très discutable et très commentée par toute la filière. Ainsi, comme souvent, mes chers collègues, il aura fallu deux événements majeurs pour que nous nous rendions compte de la triple chance qu'avait notre pays de disposer d'une énergie à un coût relativement bas,

Le discours du Président de la République, qui souhaite que la France investisse 1 milliard d'euros dans l'énergie nucléaire d'ici à 2030, avec la construction de petits réacteurs, va dans la bonne direction. pouvait bien évidemment pas suffire ... Si, d'un côté, la politique du mix énergétique doit être poursuivie, avec bien sûr la montée en puissance des énergies renouvelables, de l'autre, la France doit impérativement renouveler son parc de réacteurs nucléaires. Ainsi, la semaine dernière, M. Emmanuel Macron a annoncé vouloir mettre en oeuvre un nouveau plan pour le développement du nucléaire dans les prochaines années.

de soutien à l'excellence de la filière. Le reste des modalités sera annoncé prochainement et soumis à débat public. Il ne m'appartient pas de faire des annonces ici, aujourd'hui, mais les orientations générales sont bien celles répartition dans le temps des fermetures programmées des réacteurs arrivant en fin de vie, pour éviter l'effet falaise ; développement du nouveau nucléaire sur base d'EPR et de SMR ; enfin, soutien à l'innovation, à la technologie et à l'excellence. Il s'agit des fondamentaux du volet nucléaire de notre stratégie et de notre souveraineté énergétiques.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je vais essayer de résumer la position de notre commission des affaires économiques, qui, comme vous le savez, est très attachée à la souveraineté énergétique. Comme l'a souligné notre collègue Serge Babary, une énergie peu chère et peu émissive conditionne tout à la fois le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité des entreprises et la décarbonation de nos modes de production et de consommation. C'est la condition pour une économie résiliente, capable de soutenir la concurrence, de s'insérer dans la mondialisation et de tirer profit de son ouverture, plutôt que d'en subir les contrecoups, comme aujourd'hui. Or, si notre souveraineté énergétique a longtemps semblé aller de soi, en raison de la force de l'énergie nucléaire, la diversification de notre mix la met aujourd'hui incontestablement au défi. Que l'on en juge : tout d'abord, la filière économique, malgré les annonces, est toujours en berne. La loi de transition énergétique de 2015 impose la fermeture de quatorze réacteurs nucléaires, les deux réacteurs de Fessenheim ayant cessé de fonctionner en mars et en juin 2020 ; Mme Pompili connaît bien cette décision, dont elle a été actrice lors du précédent quinquennat. Dès lors que ces réacteurs sont viables sur le plan de la sûreté nucléaire, de tels arrêts sont un immense gâchis, une perte de valeur, un non-sens au regard de nos objectifs énergétiques et climatiques. Tout à fait ! C'est la raison pour laquelle notre commission a allongé le calendrier de fermeture de dix ans dans la loi Énergie-climat de 2019. Elle a, en outre, conditionné toute nouvelle fermeture de réacteur à une étude d'impact sur la sûreté nucléaire, sur la sécurité d'approvisionnement et sur nos émissions de CO2 dans la loi Climat et résilience de 2021. Pis, au-delà du parc existant, les perspectives de construction de réacteurs de troisième génération ou de recherche sur ceux de quatrième génération le souligner, mes chers collègues. Si la construction de nouveaux réacteurs a été annoncée, on ne sait rien de concret sur leur nombre, leur type, leur coût, le calendrier, alors que la durée minimale d'un chantier est de dix ans- quinze ans, disiez-vous, madame la ministre -et que le parc actuel fera face à un effet falaise dès 2040. Il y a donc urgence à offrir de la lisibilité aux industriels, mais aussi aux citoyens et aux parlementaires. Par ailleurs, les projets de recherche nucléaire ne sont pas assez soutenus. Je pense naturellement au démonstrateur de réacteur à neutrons rapides Astrid, projet abandonné en 2019 et pourtant prometteur pour réussir la fermeture du cycle du combustible. Madame la ministre, c'est une faute ! Je pense aussi au réacteur à fusion d'hydrogène ITER, que la France peut s'enorgueillir La nécessité de renverser cette situation a été rappelée dans notre résolution, adoptée par le Sénat en mars dernier. Je rejoins la position de notre collègue Gérard Longuet : la reconnaissance du nucléaire dans la taxonomie européenne est indispensable, mais elle est mal engagée- vous le savez, madame la ministre. C'est d'ailleurs le signe d'un manque d'influence de notre pays au sein de l'Union européenne. Hormis l'énergie nucléaire, les filières des énergies renouvelables sont insuffisamment valorisées. Si je me réjouis que le Premier ministre ait indiqué, cet été, que « la croissance verte s'appuie sur l'hydroélectricité », tel n'a pas toujours été le cas. Il ne fut pas simple, cher Daniel Gremillet, de faire aboutir notre proposition de loi sur l'hydroélectricité, adoptée à l'unanimité du Sénat en mars dernier, puis intégrée à la loi Climat et résilience en août. Pourquoi une telle hostilité à l'égard de cette source d'énergie renouvelable, la plus ancienne, la plus importante et la plus territorialisée ? Par ailleurs, l'essor légitime et nécessaire des énergies renouvelables ne doit pas détériorer notre souveraineté énergétique. Or ces énergies ont une face sombre : leur dépendance aux métaux rares. C'est pourquoi il faut favoriser non seulement la production d'équipements, mais aussi l'extraction de métaux en France et en Europe. Dans la loi Énergie-climat de 2019, la commission a donc appliqué le critère du bilan carbone aux projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres. Elle a prévu son extension aux projets attribués en guichets ouverts et a consacré un objectif de souveraineté minière dans la loi Climat et résilience de 2021. Nous attendons du Gouvernement qu'il réponde réellement et concrètement aux enjeux posés par notre souveraineté énergétique. Pour ce faire, il doit revaloriser l'énergie nucléaire, consolider les énergies renouvelables et, corrélativement, veiller au projet minier, la souveraineté minière étant au fondement de notre souveraineté énergétique. La loi quinquennale prévue en 2023 doit poser les concours de cette reconquête énergétique,

J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et de la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques sont parvenues à l'adoption de deux textes communs.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dissipons tout malentendu : à partir du 1 janvier prochain et pour six mois, la France ne présidera pas l'Union européenne, mais assumera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. de l'une des quatre institutions européennes majeures, puisqu'elle adopte la législation européenne avec le Parlement européen et développe la politique étrangère et de sécurité de l'Union, selon les orientations du Conseil européen.

ainsi, l'Allemagne et la Finlande ont échangé leur présidence, en 2006, pour cause d'élections législatives. La France n'a rien demandé de tel. Le Président de la République a donc souhaité cette présidence, qu'il veut faire coïncider avec les derniers mois de la sienne. C'est un exercice périlleux, politiquement tout d'abord. d'abord. Il l'est au premier chef pour les membres du Gouvernement, qui devront assurer la présidence des différentes formations du Conseil- sauf vous, monsieur le ministre, puisque le conseil Affaires étrangères reste présidé par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Naturellement, dans le sillage du Gouvernement, le président français se trouvera valorisé sur la scène européenne, même s'il ne présidera pas le Conseil européen, dont la présidence stabilisée est aujourd'hui confiée à Charles Michel. Le risque de confusion, en période électorale, est évident. Cette présidence compressée est aussi un exercice périlleux pour notre pays, car l'expérience montre que l'imprévu s'invite toujours à la table européenne. On l'a vu en 2008, lorsque notre dernière présidence a été bouleversée par la crise financière. La crise sanitaire représentera déjà un défi énorme, mais d'autres crises pourraient survenir, se cumuler et, finalement, accaparer notre semestre de présidence. Lorsque la commission que je préside a auditionné le secrétaire général des affaires européennes et le secrétaire général de la présidence française, voilà un an, je me suis inquiété de savoir comment notre pays pouvait mener de front la gestion d'une crise au niveau européen et une campagne électorale présidentielle, puis législative, au niveau national.

Je comprends, monsieur le ministre, que le Gouvernement entend s'en remettre aux fonctionnaires pour assumer la présidence au deuxième trimestre. Mais reconnaissez que ce n'est pas satisfaisant. Il ne nous reste plus qu'à espérer que les crises ne seront ni trop nombreuses ni trop Une présidence du Conseil, c'est aussi un exercice contraint. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux commencés de nombreux mois, voire de nombreuses années auparavant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les présidences fonctionnent en trio : en l'occurrence, la présidence française ouvre les dix-huit mois d'un nouveau trio associant notre pays à la République tchèque et à la Suède, qui lui succéderont. Nous devrons convenir d'une programmation de moyen terme, dans laquelle inscrire notre propre programme semestriel de court terme. Si Si la présidence se doit d'être neutre et de rechercher avant tout un compromis dans l'intérêt général européen, elle joue aussi un rôle d'impulsion, ne serait-ce que par la maîtrise du calendrier et de l'ordre du jour. C'est sur ces priorités que nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui. Voilà un an, le Gouvernement a annoncé que la présidence française serait construite autour de trois mots-clés : relance, puissance, appartenance. Puis, il a constitué un comité de réflexion et de propositions pour donner au travail technique et législatif une cohérence d'ensemble, en intégrant la diversité des enjeux. la commission des affaires européennes a entendu le président de ce comité, M. Thierry Chopin, ainsi que trois autres de ses membres. Je reconnais que la réflexion qu'ils avaient engagée semblait prometteuse. Elle devait aboutir cet automne. Où en est-elle ? Espérons que vous nous en direz plus, car nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'échéance. Dans cette attente, nous tenions à attirer votre attention sur les enjeux que le Sénat juge majeurs pour ce prochain semestre. Il s'agit tout d'abord de la relance, car il est essentiel de consolider la sortie de crise après le choc profond de la pandémie. Le plan de relance se décline partout en Europe, son financement par l'emprunt est acquis, mais la France devra faire avancer la discussion sur les ressources propres de l'Union européenne, car elles en sont la contrepartie indispensable. Nous fêterons aussi en janvier prochain les vingt ans de l'euro, et cela doit nous conduire à examiner son bilan pour consolider son avenir, également comme monnaie numérique. Il importera aussi d'ouvrir des perspectives nouvelles au service de la finance et du capitalisme responsables, sans oublier le devoir de diligence des entreprises et la mise en place d'un salaire minimum. Ensuite, l'autonomie stratégique se construit bien sûr en matière de défense. L'affaire des sous-marins nous l'a cruellement rappelé l'Europe doit pouvoir compter sur ses propres forces. Le haut représentant Josep Borrell l'a confirmé hier, en vous présentant, ainsi qu'à vos vingt-six homologues, la « boussole stratégique » de l'Union, qui vise à la création d'une capacité autonome de déploiement rapide. Le moment est propice. Très structurante pour notre sécurité et notre résilience, la boussole devra être finalisée en mars 2022, pendant la présidence française. Sans doute notre pays devra-t-il pour cela éviter le discours de la puissance, qui raidit nos partenaires, mais assurément favoriser une affirmation de l'Union européenne comme centre de pouvoir ouvert. Cette affirmation, notre présidence devra également la défendre à l'égard du Royaume-Uni. L'autonomie stratégique se construit aussi sur le plan technologique : l'Europe doit remédier à ses vulnérabilités structurelles, dans des secteurs clés comme la santé, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et bien sûr le spatial. Conclure les négociations sur les actes régulant les marchés et services numériques s'impose aussi comme un objectif décisif de notre présidence, car il s'agit d'affranchir l'Europe de sa dépendance aux Gafam. L'enjeu est le même en matière d'indépendance énergétique. Aussi la France doit-elle veiller à obtenir l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie des investissements verts. Nous venons d'avoir un débat sur ce sujet. Tenez-en compte,

aussi bien dans la Manche que dans le contexte des attaques hybrides que mène la Biélorussie sur la frontière orientale de l'Union et de l'effondrement de l'Afghanistan. La négociation du pacte européen pour l'asile et les migrations est gelée, et notre pays aura la responsabilité de trouver une issue pour la redynamiser, au service d'une sécurisation des frontières européennes et d'une plus grande solidarité avec les États de première entrée. Néanmoins, il devrait aussi - je reviens d'Italie avec cette conviction encourager la Commission à travailler sur la dimension extérieure de ce sujet et à nouer des partenariats avec les États de départ, notamment africains, en capitalisant sur leur relation avec certains États membres. Dernier défi à relever : nourrir nourrir l'appartenance. Cela passe non seulement par un dialogue sur le sens que les Vingt-Sept donnent aux valeurs qui les unissent et sur l'identité de l'Europe, questionnée par le Brexit et les partisans de l'élargissement aux Balkans, mais aussi par la promotion de la culture européenne et du multilinguisme et par une réflexion sur le moyen d'articuler la primauté du droit européen et le respect de l'identité constitutionnelle des États membres. Sur l'ensemble de ces sujets, la Conférence sur l'avenir de l'Europe avancera sans doute des propositions au printemps. Veuillez conclure, mon cher collègue. Notre pays sera-t-il alors en mesure de les recevoir ? Pour sa part, le Sénat, qui sera tout au long du semestre la seule institution stable de notre République,

l'urgence climatique, le durcissement de la vie internationale et les inconnues de la révolution numérique ? À mes yeux, la réponse est très claire : ces bouleversements globaux sont autant de défis que nous ne pouvons espérer relever pleinement que si nous y faisons face en Européens, avec nos partenaires des Vingt-Sept à nos côtés. C'est la conviction qui a toujours guidé l'action du Président de la République et du Gouvernement. C'est pourquoi la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui commencera le 1 janvier prochain, constitue, pour nous, une échéance politique décisive. Alors que nous entrons dans la toute dernière ligne droite, je me réjouis de pouvoir évoquer avec vous les avancées de notre travail de préparation, dont il reviendra au Président de la République de présenter aux Français les premières orientations, au début du mois prochain. Ce que je puis d'ores et déjà vous indiquer, c'est que l'impératif de souveraineté européenne, que vous avez évoqué, monsieur le président de la commission, avec l'autonomie stratégique, sera notre fil d'Ariane pour accélérer le vaste mouvement de prise de conscience qui parcourt l'ensemble de notre Europe depuis qu'elle a commencé à sortir à sortir du temps de la naïveté et de l'innocence pour ouvrir pleinement les yeux sur les formes de dépendance excessive dans lesquelles nous avons pu nous laisser entraîner, sur la brutalisation du monde et sur les risques de fracture menaçant notre Union. Pour répondre à chacun de ces dangers, nous devons nous mettre en capacité de faire nos propres choix, en affirmant cette souveraineté collective, qui, dans un monde de compétition à outrance, est de toute évidence le prolongement et la meilleure garantie de nos souverainetés nationales. Oui, j'y insiste : la souveraineté collective que les Européens affirment ensemble, c'est aujourd'hui le prolongement et la meilleure garantie de la souveraineté de la France ! C'est un fait géopolitique, stratégique et politique. C'est pourquoi il n'y a pas à choisir entre la France et l'Europe. Comme le disait le Président de la République, en s'adressant à nos compatriotes voilà tout juste une semaine, « la France ne sera pas forte toute seule ». Car notre Europe, en nous donnant le surcroît de puissance et d'influence qui rend notre nation plus solide et plus robuste pour affronter la mondialisation, vient consolider les forces qui sont les nôtres.

Il s'agit de rebâtir nos capacités industrielles et technologiques, en misant sur l'innovation, notamment par le lancement de nouveaux Piiec, les projets importants d'intérêt européen commun, sur l'électronique, la connectivité 5G-6G, ainsi que sur l'hydrogène. Pour réarmer l'économie européenne, nous continuerons aussi à nous battre pour que nos entreprises jouent à armes égales avec leurs concurrentes dans une économie mondialisée, en luttant contre toutes les formes de concurrence déloyale. Des textes sont en préparation ; ils devraient aboutir au cours de notre présidence. Il s'agit aussi d'avancer dans la construction de l'Europe de la santé, dont nous avons su poser les bases au coeur même de la première vague pandémique, en brisant des tabous et en allant même au-delà de nos traités. Il s'agit également de donner corps à l'idée d'une Europe sociale, qui n'est plus, désormais, un simple slogan.

plus efficacement contre les contenus illicites et préjudiciables. C'est pourquoi nous ferons tout notre possible pour faire avancer les négociations sur les règlements DMA et DSA, afin de continuer à bâtir, étape par étape, un modèle de régulation numérique européen. Il s'agit, enfin, de travailler à mettre en oeuvre le Pacte vert proposé par la Commission en juillet dernier. De la COP21, dont nous avons défendu les acquis contre vents et marées, à la COP26 qui vient de s'achever, l'Europe a souvent montré la voie. Le pacte de Glasgow pour le climat, s'il enregistre de réels progrès, montre bien que les efforts doivent se poursuivre pour que nous soyons, collectivement, à la hauteur de la situation et de sa gravité. C'est bien pour cette raison que nous continuerons à avancer, sur notre continent, par des actes concrets. Pour autant, nous veillerons également à ce que l'Union ne retombe pas dans une forme de naïveté, qui consisterait à sacrifier notre compétitivité et l'attractivité économique de notre continent. Collectivement, nous avons su faire preuve d'une détermination remarquable remarquable en nous fixant un double objectif de réduction de nos émissions d'au moins 55 % en 2030 et de neutralité climatique en 2050. Nous devons, ensemble, faire preuve de la même détermination pour nous assurer que notre politique environnementale ira de pair avec la préservation de nos intérêts et l'affirmation de règles de concurrence plus équitables au niveau international, en mettant en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes et en faisant du respect de l'accord de Paris une clause essentielle de nos accords de libre-échange. Cette souveraineté réaffirmée n'est tenable que si, dans le même temps, notre Europe assume enfin la puissance qu'elle porte en elle. Ce sera donc la deuxième ligne de force de notre présidence. Disons-le, pour des raisons qui tiennent à l'histoire dont elle est le fruit, notre Union n'a pas toujours eu le réflexe de la puissance. Pourtant, là aussi, une prise de conscience commence à faire bouger les lignes, à l'échelle du continent. En témoignent les progrès de la défense européenne, qui se poursuivront, grâce à l'adoption, je l'espère, sous présidence française, de notre première boussole stratégique, qui doit tirer toutes les conséquences du recentrement de notre allié américain sur une définition plus ciblée de ses intérêts fondamentaux.

ne pourra se faire que dans le cadre d'un rééquilibrage et d'une refondation des liens entre les États-Unis et les Européens. Et les échanges que le Président de la République et le président Biden ont eus à Rome à la fin du mois dernier montrent que notre partenaire américain commence à intégrer cette nécessité. Ce qui témoigne aussi de cette prise de conscience stratégique, c'est le regard nouveau, plus pragmatique et plus lucide, que nous portons désormais sur les atouts qui sont les nôtres : notre marché intérieur, qui est le premier marché au monde et qui constitue notre meilleure base arrière pour peser dans la mondialisation notre rang de premier bailleur mondial d'aide publique au développement ; nos efforts pionniers dans la régulation du numérique. Il s'agit non pas seulement de fiertés européennes, mais aussi, à une époque d'extension de la compétition géopolitique à tous les champs de la vie internationale, de nouveaux attributs de puissance. Et nous sommes en train de le comprendre, à vingt-sept ! Nous saisissons enfin que l'Europe est armée pour être une grande puissance du XXI siècle, à condition, mais cette condition est essentielle, que nous fassions un usage stratégique de ces atouts.

Assumer notre puissance européenne, c'est aussi construire de nouvelles voies de coopération, particulièrement dans les régions qui ont une importance stratégique au regard de nos intérêts et de ces biens communs qu'il est, au fond, également de notre intérêt de défendre. Je pense notamment à l'Indo-Pacifique et à l'Afrique.

les éléments du pacte sur la migration et l'asile puissent avancer. Vous y avez fait référence, monsieur le président de la commission. Il faut tirer toutes les conséquences des phénomènes migratoires que nous constatons, toujours dans le respect de nos valeurs, en trouvant le juste équilibre entre responsabilité des États de première entrée et solidarité de tous les États membres, ne serait-ce que pour ne plus donner prise aux instrumentalisations cyniques et aux tentatives de déstabilisation inacceptables de certains dirigeants étrangers, à commencer par M. Loukachenko.

qui entourent les actuelles tractations politiques chez notre principal partenaire, l'Allemagne, limitent encore la visibilité de ce qui pourra réalistement être engagé. À cette incertitude s'ajoute celle d'une actualité imprévisible, qui vient régulièrement bousculer un agenda européen déjà très contraint, sous la forme de crises et de tensions nouvelles appelant des réponses rapides et si possible coordonnées. Entre le devoir de répondre à ces crises impromptues et la nécessité de renforcer les fondations de l'Union, sous peine d'un déclassement international, il est d'ores et déjà indispensable de se doter d'instruments visant à prévenir des menaces qui se profilent à bas bruit, mais qui ne devraient pas manquer malheureusement de s'amplifier dans les mois à venir. Parmi ces sujets de préoccupation, la question de la protection des libertés académiques au niveau européen est loin d'être anodine. La récente mission d'information sur ce sujet, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, a mis en lumière les effets dévastateurs des ingérences étatiques extraeuropéennes dans nos universités et la nécessité de prendre des mesures pour préserver nos libertés académiques et protéger notre patrimoine scientifique. Le problème n'est pas, tant s'en faut, propre à la France. Les travaux menés par Scholars at Risk et le Global Public Policy Institute mettent clairement en lumière les menaces qui pèsent sur les libertés académiques dans la plupart des pays de l'Union, libertés qui constituent le fondement de l'indépendance, de l'intégrité et de la qualité de nos systèmes universitaires et de recherche. Pourtant, nous manquons aujourd'hui d'un cadre juridique solide à l'échelle européenne pour protéger ces valeurs essentielles. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que la présidence française pourrait être l'occasion d'accélérer l'élaboration du cadre à mettre en oeuvre dans ce domaine à l'échelle européenne ? Monsieur le sénateur André Gattolin, vous avez produit un rapport très pertinent sur les nouveaux risques qui se présentent à nous, en particulier les stratégies d'influence agressives, qui brouillent les frontières et, parfois, normalisent certaines formes d'ingérence. Vous avez souhaité, dans votre rapport, qu'il y ait une prise de conscience renforcée de ces menaces et de ces risques. J'ai coutume de dire

dans la zone indo-pacifique, où des alliés n'hésitent pas à nous livrer une concurrence acharnée au péril de nos relations. Je pense aussi à la détérioration sans précédent de la situation économique du Liban, à la crise diplomatique avec l'Algérie, aux tensions au Sahel et, plus récemment, aux agissements de la Biélorussie, qui instrumentalise une crise migratoire. Le monde bouge vite, et nous constatons toujours la lenteur des réactions de l'Union européenne. Celle-ci est due non pas à un manque d'outils ou de mécanismes pour réagir, mais à une absence de vision claire et partagée. États membres ont des histoires différentes, bien qu'elles soient communes, des ambitions diverses, bien qu'elles soient entremêlées, et l'Union n'est à son aise que dans le compromis. Pourtant, une vision ambitieuse à la hauteur de notre continent est nécessaire. C'est l'objectif, vous l'avez rappelé, de la boussole stratégique qui a été lancée durant la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Notre pays aura en charge de la finaliser. Les enjeux sont multiples, mais résident principalement dans notre rapport avec les grandes puissances mondiales. La stratégie de la Chine est complexe et efficace, surtout en Europe. De leur côté, les États-Unis ont leur propre agenda. Quant à nous, Européens, nous n'avons pas pas tous la même relation à ces pays, et notre division est une faiblesse. La crise sanitaire a été révélatrice de notre niveau de dépendance. Il est devenu primordial de nous doter d'une stratégie multidimensionnelle et globale. Monsieur le ministre, pendant la présidence française, comment comptez-vous mettre les Européens d'accord sur une boussole stratégique ambitieuse, dont vous avez reçu les plans hier, et particulièrement sur la stratégie à déployer face à la Chine et aux États-Unis ? La parole est à M. le ministre. Vous posez, monsieur le sénateur Guerriau, des questions essentielles. Vous l'avez rappelé, la boussole stratégique a été communiquée hier au ministre des affaires étrangères de l'Union européenne. Il s'agit en quelque sorte d'un Livre blanc de sécurité et de défense. C'est la première fois qu'existent, dans l'histoire de l'Union européenne, un tel document et une telle volonté.

porte sur la déclinaison de l'une des priorités de la présidence française, celle de l'autonomie stratégique, dans le domaine de la santé, plus particulièrement des produits de santé. En effet, même si les entreprises européennes n'ont pas démérité dans la course aux vaccins, la crise sanitaire a illustré le besoin de reconquête d'une plus grande autonomie à l'échelle du continent, en particulier dans l'hypothèse, avérée au plus fort de la crise, de la rupture ou de la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Le sujet est complexe, tant il est évident que nous avons intérêt à privilégier le développement d'activités innovantes à forte valeur ajoutée sur notre territoire, alors que le besoin peut aussi se faire sentir d'une production industrielle portant sur des produits moins élaborés. C'est donc la question de la flexibilité de notre outil industriel qui est ainsi posée. La tentation est forte de faire peser cette politique industrielle sur l'assurance maladie. La sécurité sociale y prend bien sûr sa part, en solvabilisant très fortement la dépense de produits de santé. Mais elle ne peut assumer seule cette politique, qui nécessite des investissements importants. Monsieur le ministre, dans quels termes le Gouvernement entend-il porter ce sujet au niveau européen sous la présidence française ? La parole est à M. le ministre.

les premières bases d'une véritable Europe de la santé, même si celle-ci a été critiquée au début. Sans doute n'était-elle pas à la hauteur, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une compétence de l'Union européenne. Depuis lors, elle a réussi, d'une part, à mutualiser les efforts des États membres en réalisant des achats groupés d'équipements de protection et de vaccins, part, à agir d'une seule voix pour négocier avec les laboratoires pharmaceutiques au meilleur coût. Elle a également permis de lutter contre la pénurie et les goulets d'étranglement, en mettant en place un contrôle des exportations de doses, face à des partenaires et des industriels qui ne respectaient pas toujours les engagements pris et, progressivement, de faire monter en puissance la production européenne. Au cours

les mandats du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies et l'Agence européenne des médicaments. Nous ferons en sorte que ce paquet aboutisse dans le cadre de la présidence française, avec d'autres sujets, qu'il conviendra de mettre sur la table, pour nous nous doter des compétences santé les plus essentielles. J'aurais d'ailleurs l'occasion, pour la première fois, d'organiser une réunion commune des ministres des affaires étrangères et des ministres de la santé,

pour l'industrie des produits de santé, en définissant des priorités et en favorisant des investissements structurants, à la fois dans la recherche, l'innovation et le développement industriel. La

au droit européen. L'ardoise est donc loin d'être vierge ! Biodiversité, énergie, agriculture et j'en passe, les domaines concernés par des procédures d'infraction sont nombreux.

climatique : il s'agit de lutter efficacement contre les fuites de carbone en appliquant aux importations une tarification équivalente à celle qui existe sur le marché européen De cette façon, nous ferons en sorte que l'intégrité environnementale de nos efforts ne soit pas fragilisée et ne se retourne pas contre nos entreprises, tout en incitant nos partenaires étrangers à nous suivre dans cette voie : c'est une question de cohérence et d'efficacité. Bien sûr, le MACF devra être

font l'objet d'un odieux marchandage politique. D'un côté, le président biélorusse Alexandre Loukachenko instrumentalise les malheurs et les espoirs de ces migrants en les jetant sur les barbelés de la frontière polonaise après les avoir cyniquement acheminés sur place. De l'autre, le gouvernement polonais attise la haine et le racisme contre les migrants, surélève les barbelés, parle de construire un mur et envoie l'armée pour tirer si nécessaire. Ce gouvernement, qui fustige les droits humains fondamentaux, clame qu'il se moque du droit européen et sabote depuis des années toute tentative de créer une politique commune solidaire d'accueil des migrants appelle aujourd'hui l'Union européenne à se tenir à ses côtés, pour en fait l'entraîner dans la confrontation. Les surenchères vont bon train. Force est de constater que si, pour l'essentiel, elles accablent à juste titre le régime biélorusse, elles exonèrent le gouvernement polonais, qui fait maintenant appel à l'article 4 du traité fondateur

pour appliquer pleinement le respect du droit international de l'asile ? S'engagera-t-elle pour des politiques européennes s'attaquant aux causes de l'exil- les guerres, les changements climatiques et les pillages de ressources, dans lesquels les pays européens ont de lourdes responsabilités -et pour la construction de voies légales, coopératives et sécurisées de migration, seules à même de tarir les trafics humains d'exploitation de la misère

hier les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, une posture à la fois de soutien et de solidarité, parce que le but de la manoeuvre n'échappe à personne : c'est de déstabiliser l'Union européenne

Le Président de la République a récemment annoncé la relance de la création de réacteurs nucléaires. À la veille de la présidence tournante française, cette annonce me paraît bienvenue, mais elle nécessite d'être défendue En effet, faire du nucléaire une activité verte suscite de fortes réticences de la part de nos partenaires européens ; certains pays exercent notamment un intense pour écarter l'énergie nucléaire des obligations vertes que se fixe l'Union européenne dans le cadre du plan de relance. Par ailleurs, à l'heure où nous souhaitons diminuer notre consommation d'énergies fossiles, une augmentation de la part de l'électricité dans le mix énergétique, de l'ordre de 40 Le nucléaire, qui représente 67 % de notre mix électrique, est une énergie décarbonée. Sans le nucléaire, notre indépendance énergétique sera fortement remise en question, qui nous poussera à utiliser des énergies carbonées comme le gaz, en nous rendant dépendants des productions de pays qui ne sont pas forcément des démocraties. La flambée des prix de l'énergie devrait nous enjoindre à nous tourner vers le nucléaire, qui nous garantit une énergie bon marché, zéro carbone et stable.

Monsieur le sénateur, la Commission européenne s'est engagée à publier, d'ici à la fin de cette année, un acte délégué complémentaire concernant les places respectives de l'énergie nucléaire et du gaz au sein de la taxonomie verte. Ces questions ont fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières semaines. Vous le savez, l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte est soutenue au plus haut niveau politique par le Président de la République, qui s'est à plusieurs reprises exprimé sur ce sujet. Les conclusions scientifiques qui ont été rendues publiques en juillet 2021 sont globalement positives et ne font pas obstacle à l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie. une décision cohérente avec ces résultats et respectant tant le principe de neutralité technologique que la liberté des États membres de déterminer leur bouquet énergétique, liberté expressément prévue par les traités européens. Le Conseil européen d'octobre dernier a déjà été l'occasion d'aborder ce sujet entre chefs d'État et de gouvernement. Nous avons noté à ce moment-là- comme vous, j'imagine -qu'un nombre important d'États membres se sont manifestés en faveur de l'inclusion de l'énergie nucléaire dans cette taxonomie. Il est clair que le nucléaire joue et continuera à jouer un rôle important dans la réduction de nos émissions et dans la décarbonation de notre bouquet énergétique. Dans ce contexte, nous avons aussi accueilli positivement les dernières déclarations de la présidente de la Commission européenne, qui a souligné les atouts de l'énergie nucléaire et a réitéré le souhait de publier prochainement l'acte délégué complémentaire auquel je faisais référence il y a un instant. Il appartient désormais à la Commission de préciser le contenu de ces actes. Nous serons évidemment très vigilants pour que l'énergie nucléaire soit effectivement incluse dans cette taxonomie dans les prochaines semaines.

La très prochaine présidence française du Conseil de l'Union européenne ouvre une fenêtre pour insister sur ces principes, auxquels le RDSE souscrit bien naturellement. Vous y avez d'ailleurs consacré, monsieur le ministre, une large part de vos propos évoquer l'Europe de la santé, un chantier hier balbutiant, mais aujourd'hui plus prégnant, où il est en tout cas question de solidarité et de souveraineté. En effet, on a pu voir l'Europe mettre en oeuvre une réaction solidaire à la pandémie, avec l'achat en commun de vaccins, mais aussi des transferts de patients. On peut également souligner le rôle de l'Agence européenne des médicaments, qui a permis de coordonner le lancement de la campagne vaccinale, même si, hélas, tous les États membres n'avancent pas au même rythme s'agissant du taux de couverture vaccinale, avec les conséquences épidémiques que l'on constate en ce moment. Quant à la souveraineté européenne, elle ne demande qu'à s'exercer, en particulier dans le domaine de la production de médicaments et de matériel médical ; ma question portera sur ce point particulier. La pandémie de covid-19 a révélé une vraie lacune sur certains biens indispensables à la protection de nos citoyens européens, une lacune qui appelle des réponses rapides et concrètes. Dans un premier temps, on attend beaucoup de l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, mieux connue sous le sigle HERA. Quelles initiatives la France pourrait-elle prendre, dans le cadre de sa présidence, pour accélérer ce dossier ? Plus globalement, quelles seront vos priorités

Richer, que l'Union européenne avait pris à bras-le-corps l'enjeu de la santé, qui n'était pas de sa compétence, en brûlant quelque peu les étapes et les accords. Je pense qu'elle a bien fait et que les résultats ont été au rendez-vous ; maintenant, il faut les

de mettre en place HERA, la nouvelle autorité européenne qui permettra à l'UE de mieux anticiper les urgences sanitaires futures et de renforcer les circuits de recherche et de développement, d'acquisition et de distribution de contre-mesures médicales en cas de crise. Ce sera un point très important de notre présidence. Celle-ci sera aussi l'occasion d'avancer sur un autre projet important d'intérêt européen, dans le domaine des biotechnologies, ce qui permettra, en complément de l'action menée par HERA, d'aider les projets de demain qui ne peuvent aujourd'hui être développés et, ainsi, de nous maintenir à la pointe de l'innovation. Cet enjeu essentiel sera financé, puisque l'Union européenne a permis la mobilisation, dans le cadre de la politique , d'un programme de plus de 5 milliards d'euros qu'il nous faudra engager dans cette direction pour nous donner, là aussi, une forme d'autonomie stratégique dans un domaine où nous étions très absents et diminués auparavant.

elle s'impose à toutes les normes juridiques, qu'elles soient nationales ou,, d'origine européenne. Si des limitations à la souveraineté sont éventuellement admises, ce ne peut qu'être en vertu d'un consentement exprès, figurant dans la Constitution elle-même. Or, sous prétexte du prétendu principe de l'État de droit, les eurocrates veulent imposer une forme de supranationalité sans aucun fondement juridique, qui piétinerait la volonté clairement exprimée par les peuples des États membres. Voilà l'origine des conflits qui opposent l'Union européenne à la Pologne et à la Hongrie, alors que personne ne peut contester la légitimité élective des gouvernements en cause : qu'on le veuille ou non, ils ont bel et bien été élus La primauté du droit européen n'a d'ailleurs aucun fondement. En effet, comme la Pologne le souligne, cette notion ne figure dans aucun des traités de l'Union européenne. Même l'article 19 du traité sur l'Union européenne, qui sert pourtant de référence aux eurocrates, est muet sur le sujet. À l'évidence, la théorie dite « de l'État de droit » n'a donc pas à s'imposer à la volonté des peuples, telle qu'elle s'exprime lors des élections.

! Or les partisans d'une évolution de l'Union européenne vers une organisation supranationale veulent subordonner les constitutions des États membres à la dictature des eurocrates et du prétendu État de droit.

signés et ratifiés par tous les États membres, y compris la Pologne. Je voudrais aussi lui rappeler que la primauté du droit européen est un très vieux principe, qui remonte à 1964.

dans un monde marqué par une compétition internationale intense, voire par des conflictualités internationales majeures qui se jouent dans tous les domaines, à la fois sur les enjeux sanitaires, environnementaux, sécuritaires et économiques,

l'Europe est divisée, fracturée, malmenée et mal-aimée. Nous pensons qu'il faut la réparer, qu'il faut redonner confiance dans sa capacité à produire du progrès pour bâtir un monde de bien-être durable.

ni aucun territoire sur le bord du chemin. La transition écologique sera juste et inclusive ou elle ne sera pas ! La relance ne sera réussie que si elle permet un changement de paradigme économique. La seconde consiste à mettre en oeuvre les engagements des sommets de Göteborg et de Porto pour enfin construire l'Europe sociale, lutter contre les inégalités et aboutir à un salaire minimum européen. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si ces deux priorités seront, comme nous l'attendons, celles de la présidence française ? Comment, si tel est le cas, les traduirez-vous concrètement ? La parole est à M. le ministre.

des travailleurs des plateformes numériques, ainsi que leur accès à la protection sociale et au droit à la négociation collective. La Commission examine la possibilité d'une initiative dans ce domaine. Nous plaidons pour que cela soit mis sur la table pendant la présidence française. Troisièmement, enfin, la proposition législative sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes doit, elle aussi, faire l'objet d'un dépôt par la Commission, et nous voulons la faire avancer au cours de cette période. Nous souhaitons donc que l'Europe sociale progresse.

remercie, monsieur le ministre : je prends note de votre engagement, et nous aurons l'occasion, à l'issue de la présidence française, de faire le bilan des avancées. Très clairement, nous devons réorienter l'Europe et la renforcer pour mettre un terme aux souffrances des plus défavorisés et à la destruction de l'environnement. Cela passe par des avancées concrètes et rapides sur les deux priorités écologiques et sociales que nous souhaitons mettre au coeur de la Présidence française. Cela passe, plus largement, par la déclinaison du plan Climat et par la mise en oeuvre du fonds pour une transition juste, par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont nous avons parlé,

la présidence slovène en cours a porté une attention particulière aux pays des Balkans occidentaux et à leur avenir européen. Cette priorité a abouti concrètement à l'organisation du sommet occidentaux du 6 octobre dernier, qui a permis aux États membres de réaffirmer leur engagement vis-à-vis du processus d'élargissement, de renforcer la coopération dans la lutte contre le coronavirus et d'assurer le soutien à la reprise économique dans la région.

Il s'agit pourtant d'une région stratégique pour l'Union européenne et pour la France, une région qui présente d'importants enjeux en matière d'économie, de migrations et de sécurité. Des efforts de long terme sont donc nécessaires, d'un point de vue national comme européen.

Madame la sénatrice, vous savez que nous avons obtenu, il y a peu de temps, une réforme en profondeur de la méthodologie du processus d'adhésion. repose désormais sur trois principes : la progressivité, à savoir une association graduelle aux politiques de l'Union, avec des bénéfices concrets immédiats pour les populations concernées, avant même qu'il y ait un accord général ; la conditionnalité, avec un haut degré d'ambition, en particulier sur les standards et les normes, d'État de droit, un sujet particulièrement sensible dans la région à laquelle vous faites référence ; enfin, la réversibilité, qui est une condition de la crédibilité du processus, puisqu'elle permet de revenir en arrière si cela n'avance pas bien.

notre relation avec les Balkans occidentaux ne peut se résumer à la perspective de l'élargissement, en particulier dans une région soumise à beaucoup de stratégies d'influence, voire d'ingérence. Nous devons donc parallèlement promouvoir

La France assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1 janvier 2022 ; à ce titre, elle doit jouer un rôle moteur pour que les États membres ratifient, puis appliquent, les dispositions de cette convention. La France devrait être le neuvième pays à ratifier cette convention, mais cette ratification est suspendue dans l'attente d'une nécessaire autorisation européenne. Des négociations sont-elles envisagées pour faire aboutir cette décision, afin de permettre une ratification plus massive de cette convention par les États membres ? La France montrera-t-elle l'exemple pour que cette convention soit mise en oeuvre de façon ambitieuse et que les États membres ratifient, puis appliquent, les dispositions de la convention n° 190 dans des délais raisonnables ?

Face aux arguments touchant principalement aux finances, à l'environnement et aux conditions sanitaires qui nous ont été opposés de manière fallacieuse et ne résistent pas à une analyse objective, comment comptez-vous vous inscrire pleinement dans un axe fort, celui de l'esprit européen de Strasbourg, de même que dans la ligne des traités européens qui consacrent Strasbourg comme siège du Parlement européen ? La parole

évoqué la ratification de la convention de l'OIT relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Il s'agit bien d'une priorité politique pour la France, qui s'inscrit dans la grande cause du quinquennat,

car, au-delà de ce texte, l'Union européenne est une union de valeurs. Elle a développé un acquis très important dans ce domaine depuis plusieurs décennies, acquis qui a permis aux États de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sera également un sujet essentiel de notre présidence, car nous savons que le consensus indispensable

Un tel débat aurait pu avoir lieu au long cours, sur plusieurs mois, afin de nous permettre d'avancer tous ensemble : l'exécutif, la représentation nationale et les citoyens. La présidence de l'Union européenne par l'un de ses pays fondateurs aurait pu être l'occasion d'une puissante initiative pour relancer l'Union. Je fais partie de ceux qui croient à l'Union européenne non pas seulement par principe, mais parce que, plus que jamais, elle constitue un projet de construction positif dans un monde et des sociétés traversés par les menaces et les replis. À l'heure où les superpuissances sont de retour sur la scène internationale, où est la superpuissance européenne ? Comment des responsables rationnels peuvent-ils imaginer que la fermeture de frontières et rendre ces dernières infranchissables ? Comment peuvent-ils à ce point rester sourds et aveugles à l'état du monde ? La souveraineté la plus importante, c'est celle des peuples, non celle des représentations fantasmées et nationalistes, qui ne conduisent qu'au rejet et à la xénophobie. Le rejet comme norme : nous savons où un tel projet conduit inéluctablement. L'Union européenne est l'une des seules voies de recours crédibles en matière de protection internationale. Alors que nous pensions la paix acquise, celle-ci est plus que jamais menacée. Les événements ne cessent de nous rappeler sa fragilité. Certes, Certes, le président Mitterrand nous avait prévenus, lui qui appelait à toujours s'engager davantage dans le processus de construction européenne. Alors que la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union, le silence règne : rien ou presque. Deux sujets sont majeurs pour l'avenir proche de l'Europe et de l'ensemble de nos pays au sein de l'Union : la diplomatie et la défense. Vous avez évoqué, monsieur le ministre, l'Europe de la défense. Aussi, voici ma question : quelles mesures réelles la France entend-elle prendre durant sa présidence pour accroître l'intégration des membres de l'Union en matière de défense et de diplomatie ? Où en est-on, par exemple, des projets de système de combat aérien du futur, après les atermoiements de l'Espagne

est à M. Cyril Pellevat. Monsieur le ministre, la présidence française du Conseil de l'Union européenne approche à grands pas. Je pense que nous partageons tous le souhait qu'elle soit l'occasion d'avancer sur plusieurs dossiers d'une importance capitale pour l'Europe et la France, tels que la relance économique, le pacte sur la migration et l'asile, la transition écologique ou encore la régulation et la sécurité en matière de numérique. C'est sur ce dernier point que j'insisterai, notamment sur la question de la cybersécurité. (RGPD) a été un véritable modèle dans le monde en matière de protection des données. Je pense qu'il est aujourd'hui temps que l'Union européenne soit de nouveau un moteur sur un sujet d'une importance capitale : la cybersécurité. Bien évidemment, la cybersécurité est un sujet relevant de la souveraineté des États, plus particulièrement de leur souveraineté numérique.

Une première étape a été franchie avec la directive (NIS), puis une nouvelle avec la stratégie de cybersécurité de l'Union européenne et la création de l'unité conjointe de cybersécurité, mais nous devons aller plus loin et tendre vers des souverainetés numériques individuelles, qui soient interopérables.

Ainsi, en fluidifiant les interactions, une réelle puissance européenne en matière de cybersécurité pourrait se construire, sans transfert de souveraineté. L'Union européenne pourrait être un véritable leader en la matière, en fixant des standards qui auraient alors une répercussion mondiale. est donc, monsieur le ministre, la position du Gouvernement sur ce sujet ? Est-il prévu de légiférer sur la question de la fixation de standards et de critères européens en matière de cybersécurité et sur l'interopérabilité des souverainetés numériques des États au cours de la présidence française du Conseil ? La parole

vous posez des questions tout à fait opportunes sur un enjeu essentiel de souveraineté. J'adhère tout à fait au concept de souveraineté numérique. Durant la présidence française, nous accélérerons l'examen d'une série de propositions qui sont déjà sur la table.

mène aussi des actions contraires au droit européen à cette même frontière. Il est terrible, monsieur le ministre, de constater que, face à une menace commune, il existe des gouvernements en Europe

Pour éviter ce type de comportement de la part d'États membres, il convient, monsieur le ministre, de conférer une légitimité démocratique plus forte aux politiques européennes.

? En outre, cela a été dit, nous connaissons actuellement de nouveaux phénomènes migratoires, du fait notamment de la crise afghane, dont on n'a pas encore mesuré les conséquences probables, et de l'afflux de migrants arrivant par la Biélorussie.

difficilement atteignables, parce que chaque État concerné verra uniquement ses propres intérêts. Je ne vois pas comment on pourrait faire passer le paquet asile-migration dans un tout.

Nous devons peut-être aussi renforcer le contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne en instaurant des procédures frontalières efficaces, là encore de manière pragmatique. Enfin, sur ce dernier point, je pense que nous devrions pouvoir avancer plus vite que sur les autres et alléger la pression à nos frontières en intensifiant notre coopération avec les pays d'origine et de transit,

Bien qu'elle soit au centre des discussions politiques à Bruxelles, elle n'a toujours pas permis à ce jour de résorber les écarts socio-économiques entre régions européennes. Les phénomènes, pour ne pas dire les stratégies assumées, de dumping social qui en résultent minent non seulement l'efficacité du marché unique, mais aussi, et surtout, la confiance de nos concitoyens, qui attendent d'abord de l'Europe qu'elle les protège. Certes, plusieurs mesures concrètes en matière de convergence sociale européenne ont été engagées récemment, mais elles restent à ce stade très légères. dans l'Union européenne, qui avait suscité de grandes attentes, est finalement décevante, sa portée étant trop limitée. Quant au plan d'action pour la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux, il repose presque en totalité sur la bonne volonté des États membres, dont certains restent réticents à toute idée de convergence sociale. Monsieur le ministre, vous avez affirmé que la présidence française de l'Union européenne porterait une ambition sociale forte.

car elle permettra de garantir des droits fondamentaux, en particulier celui de vivre de son travail. Nous aurons à coeur de faire avancer ce sujet sous la présidence française. Un compromis est désormais envisageable,

et, d'une certaine manière, de la pérennité du projet européen. Si nous arrivons à faire aboutir ce texte, nous aurons fait un pas en avant considérable. Je ne pense pas utile de remettre aujourd'hui sur la table la directive sur les travailleurs détachés,

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a mis en exergue l'importance de la sauvegarde du patrimoine de proximité, des campagnes et des petites villes, telles que les petites cités de caractère, qui forment un cadre de vie dans lequel une part croissante de nos concitoyens aspirent à vivre. Un nouvel exode urbain vers les campagnes à l'oeuvre. La conservation et l'animation culturelles, entre autres, sont des atouts non négligeables, non seulement pour la préservation d'un cadre de vie de qualité, spécifiquement européen, mais aussi pour l'attractivité économique. Cette question de civilisation et d'identité culturelle européenne peut-elle faire partie, monsieur le ministre, des priorités de la présidence française ? Monsieur le sénateur, vous avez tout à fait raison de soulever cet enjeu, d'autant plus que la culture a durement pâti de la pandémie et qu'elle en reste affectée. C'est un enjeu clé qui parle à nos concitoyens. La culture suscite un sentiment d'appartenance européenne. Il importe donc de cultiver cette dimension. Dans ce contexte, nous agirons agirons dans trois directions. Tout d'abord, nous contribuerons à faire vivre la culture européenne par l'organisation de manifestations en France et dans le monde. Ainsi, nous organiserons une Nuit européenne des idées, qui permettra de souligner le rôle de la France comme passeuse de culture au sein de l'Union. Tout notre réseau diplomatique et culturel sera mobilisé pour que cet événement rayonne dans le monde. Nous organiserons aussi la Fabrique Europe au Grand Palais, qui accueillera au début du mois de février six cents jeunes Européens, professionnels de la culture et des arts, et deux cents professeurs. Ils seront invités pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe et réaliser des oeuvres en lien avec les symboles de l'Europe. Ils formeront ainsi un réseau européen de créateurs. De nombreux événements seront également consacrés à la promotion de la diversité culturelle et linguistique, afin de souligner l'importance du multilinguisme et de promouvoir l'usage du français, notamment dans les institutions européennes. Ensuite, nous essaierons de faire avancer l'agenda de souveraineté européenne de souveraineté européenne d'un point de vue culturel et nous veillerons à ce que les avancées qui ont été obtenues récemment grâce à la directive sur le droit d'auteur, qui permet de protéger, donc de stimuler, la création, ou à celle sur les services de médias audiovisuels, qui permet de garantir la diffusion de 30 % d'oeuvres européennes sur les plateformes, soient bien mises en oeuvre. Il s'agit d'avancées considérables, en faveur desquelles, vous le savez, notre pays s'est beaucoup mobilisé. Enfin, nous mettrons l'accent sur les enjeux du patrimoine, car notre politique en

Il a montré combien l'attente du Sénat était grande envers cette présidence. Ce débat a également permis de soulever les nombreuses incertitudes qui entourent déjà notre présidence, avant qu'elle ne débute : la nouvelle flambée épidémique, les transitions politiques à l'oeuvre dans plusieurs États membres, mais aussi dans le voisinage de l'Union, la pression migratoire, qui s'exerce chaque jour un peu plus fortement à nos frontières, les tensions géopolitiques croissantes, y compris au coeur du continent européen. Dans cette mer agitée, l'Union aurait grand besoin d'une boussole stratégique, mais celle-ci n'est pas encore finalisée, et d'un capitaine, mais le Président de la République du pays chargé de la présidence pourrait bien changer au milieu du gué. Nous pouvons légitimement être inquiets. L'Union aurait surtout besoin que soit fixé un cap à long terme. Plusieurs collègues l'ont souligné, l'Europe a besoin de trouver les moyens de s'affirmer auprès des Européens et de ses partenaires internationaux. Elle s'est justement lancée dans un exercice d'introspection. La Conférence sur l'avenir de l'Europe a enfin été lancée en mai dernier, sur une idée du président Macron, reprise par la présidente de la Commission européenne. Cet exercice de démocratie directe vise à dégager des orientations pour consolider durablement le projet européen. Il mobilise beaucoup d'énergie de la part des citoyens qui siègent à son assemblée plénière ou qui contribuent sur la plateforme numérique, mais aussi de la part des parlementaires nationaux et européens qui y participent. Or la Conférence sur l'avenir de l'Europe est censée aboutir sous présidence française. À ce sujet aussi, nous sommes inquiets. Comment notre pays, focalisé sur ses élections intérieures, sera-t-il capable d'accueillir les propositions structurantes que cette conférence devrait avancer ? Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que, malgré son calendrier interne, la France ne laisse pas passer cette occasion fondamentale de remettre l'Union européenne sur les rails lui permettant de rester la plus grande démocratie du monde. Nous en

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relatives aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (projet

Le 3 août 2019, une collectivité nouvelle est née : la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). Sa création est le fruit d'un travail étroit avec ce territoire, mené afin de répondre à des enjeux spécifiques. Elle est la concrétisation de la politique de différenciation territoriale qui a été portée depuis le début de ce quinquennat et qui s'est traduite dans cette ordonnance par l'attribution à cette nouvelle collectivité de compétences spécifiques, en lien avec sa situation historique et géographique particulière. Afin de répondre aux enjeux de transport transfrontalier qui marquent ce territoire, il a été décidé de transférer le réseau routier national à la CEA et, sur son périmètre, à l'Eurométropole de Strasbourg. Après de longs mois d'échanges et de consultations, en lien avec la collectivité, des ordonnances ont été prises en mai dernier, comme le prévoyait l'article 13 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA.

Créée par la CEA, cette taxe sera versée par les usagers de poids lourds, afin de maîtriser le trafic routier sur les axes relevant de la CEA et de limiter les nuisances dues au trafic de transit des poids lourds, qui s'est reporté vers l'Alsace depuis l'instauration, côté allemand, de la .

Elle prévoit notamment un avis obligatoire du préfet sur tout projet de modification des autoroutes, afin de garantir que les aménagements envisagés par la collectivité soient compatibles avec les nécessités liées aux transports exceptionnels ou à la défense nationale, par exemple. Enfin, une ordonnance précise les conditions dans lesquelles l'Eurométropole de Strasbourg reprend les engagements de l'État vis-à-vis du concessionnaire de l'autoroute A355, appelée aussi « Grand contournement ouest de Strasbourg », dans le cadre de sa mise en service. C'est l'article 3 qui vise à ratifier cette

Les ordonnances soumises à votre assemblée pour ratification ont été rédigées dans le respect des spécificités de ce territoire, et d'importantes marges de manoeuvre lui sont laissées. C'est le cas, par exemple, sur l'instauration même de la taxe,

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a souhaité apporter plusieurs modifications à ce texte. Certains amendements visent à améliorer le dispositif. Le gouvernement partage cette ambition. à l'amendement tendant à permettre de s'acquitter de la taxe sans recourir à un équipement embarqué. Le Gouvernement y est favorable, et je sais que cet avis est partagé par la CEA. Quelques modifications techniques ou rédactionnelles pourraient toutefois s'imposer pour instaurer cette nouvelle possibilité de paiement.

Toutes ces modifications sont précieuses, même si leur rédaction nécessitera peut-être des ajustements ou des précisions après analyse juridique fine dans la suite du processus législatif.

Toutefois, d'autres modifications pourraient nuire à l'équilibre du texte, voire contrevenir au principe de libre administration des collectivités locales, auquel vous êtes, comme moi, particulièrement attachés. L'article 1 , introduit par la commission, encadre la liberté d'action de la CEA en matière de modulation de la taxe en fonction de critères environnementaux au-delà de ce qui semble à la fois nécessaire et opportun.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est singulier, à tous égards. Sur Sur la forme, tout d'abord, nous avons à discuter d'un projet de loi de ratification des trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la CEA. Outre le Outre le recours accru aux ordonnances dans la période récente, le dernier bilan annuel de l'application des lois, réalisé par notre collègue Pascale Gruny, relevait que l'écrasante majorité des ordonnances ne sont pas ratifiées dans des conditions permettant au Parlement de débattre des mesures qu'elles instituent. En conséquence, et dans le prolongement de la résolution adoptée par le Sénat le 1 juin 2021, sur l'initiative du président Larcher, je me réjouis de l'inscription à l'ordre du jour de ce projet de loi de ratification, qui permet au Parlement de se prononcer pleinement dans un domaine entrant dans son champ de compétences, en l'occurrence celui de la régulation du transport routier de marchandises et de la gestion du patrimoine routier par la Collectivité européenne d'Alsace. Sur le fond, également, ce projet de loi est particulier. Particulièrement sensible, il s'inscrit dans une histoire très mouvementée. Nous avons tous en tête le déroulé de ce que l'on pourrait appeler « le feuilleton de l'écotaxe », commençant par l'adoption, en 2006, d'une expérimentation pour mettre en place une taxe sur le transport routier de marchandises en Alsace, puis sa généralisation, en 2008, à l'ensemble du pays, jusqu'à son abandon, en 2014, sur fond de contestation, notamment bretonne. À ce jour, donc, aucune réponse concrète n'a pu être apportée à l'Alsace, qui subit pourtant des reports significatifs de poids lourds depuis 2005, année de la mise en place outre-Rhin d'une taxe sur les véhicules de transport routier de marchandises. De ce fait, certains axes, notamment le sillon rhénan, sont particulièrement congestionnés. C'est le cas de l'A35, qui, au nord de Strasbourg, est traversée chaque jour par près de 14 000 poids lourds. Cette situation entraîne des coûts substantiels d'entretien de l'infrastructure routière, mais également d'importantes externalités négatives pour l'ensemble des riverains et autres usagers de la voirie, qui sont confrontés à des problèmes de pollution de l'air, de nuisance sonore, de congestion ou encore d'insécurité. Dans ce contexte, le transfert au 1 janvier dernier à la CEA et à l'Eurométropole de Strasbourg de la propriété des routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur leurs territoires respectifs, est une avancée qu'il faut saluer. C'est une nouvelle étape de décentralisation et de mise en cohérence de la CEA et de en cohérence de la CEA et de l'Eurométropole de Strasbourg avec leurs réalités territoriales. Les trois ordonnances que le présent projet de loi tend à ratifier offrent les outils nécessaires pour accompagner ce transfert de la gestion de l'infrastructure routière. La première d'entre elles répond à une demande ancienne de l'Alsace et des Alsaciens. Elle donne à la CEA la possibilité de mettre en place, dans les six prochaines années, une taxe sur les poids lourds empruntant certains axes de son réseau routier. L'objectif est triple : compenser la dégradation de la voirie, dans une logique d'utilisateur-payeur réduire l'impact environnemental du transport de marchandises ; enfin, rééquilibrer les flux de camions en transit. L'ordonnance laisse d'importantes marges de manoeuvre à la CEA, qui sera libre de définir les catégories de véhicules taxables, le périmètre du réseau taxable, les taux kilométriques, ainsi que les éventuelles réductions et exonérations, dans le respect du cadre fixé par la directive européenne Eurovignette. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est montrée favorable au dispositif proposé, plus particulièrement à l'équilibre proposé entre la latitude accordée à la CEA dans la mise en oeuvre de sa taxe et le respect du cadre européen. Cependant, avec la commission des lois, elle a cherché à améliorer les textes suivant trois axes. Le premier axe est celui du renforcement de l'efficacité du dispositif,

La taxe alsacienne pourrait donc servir de modèle aux futures taxes régionales et être un laboratoire d'expérimentation au bénéfice des autres collectivités territoriales et de l'État. Dans ce contexte, il est indispensable que ce modèle soit particulièrement robuste et aisément transposable à d'autres territoires. C'est pourquoi la commission a cherché à renforcer son efficacité, par exemple en élargissant les marges de manoeuvre de la CEA ou en complétant la palette des solutions technologiques que celle-ci pourra mettre en place pour la constatation de la taxe. La commission a également amélioré le droit d'information de la CEA par l'État et clarifié le calendrier de ses délibérations pour la mise en oeuvre de la taxe. Suivant cette même logique, et en lien étroit avec la commission des lois, a élargi les modalités de contrôle du respect de la taxe, en donnant à la CEA la possibilité de mettre en place des dispositifs de contrôle automatisés. Enfin, elle a cherché à améliorer l'efficacité des mesures de sanction en assouplissant le dispositif proposé et en renforçant le caractère dissuasif des sanctions en cas de manipulation des équipements électroniques embarqués ou de falsification de documents. Le second axe d'amélioration repose sur une prise en compte des préoccupations des collectivités territoriales limitrophes, par la concertation et l'évaluation. En effet, la commission n'est pas restée sourde aux inquiétudes des collectivités limitrophes, qui sont préoccupées par des possibilités de report de trafic sur leurs voies et par l'articulation qui devra être trouvée entre la taxe alsacienne et de futures potentielles taxes régionales. C'est pourquoi elle a complété le texte par de nouvelles dispositions visant à créer les conditions d'une concertation entre les acteurs publics locaux, par l'intermédiaire d'un comité appelé à se réunir annuellement, jusqu'à la mise en oeuvre de la taxe, pour échanger sur la taxation des poids lourds. Elle a également renforcé les exigences d'évaluation des reports de trafic sur les voies des collectivités voisines de la CEA. Le troisième et dernier axe de progrès défendu par la commission consiste en une anticipation des évolutions du cadre européen. Attentive à ce que les délibérations de la Collectivité européenne d'Alsace ne soient pas remises en cause, dans un avenir proche, par la révision prochaine de la directive Eurovignette, la commission a permis à celle-ci d'adapter son dispositif aux futures évolutions du cadre européen, pour faire en sorte que la taxe puisse prendre en compte les évolutions des véhicules

La troisième et dernière ordonnance que le projet de loi vise à ratifier porte sur la reprise, par l'Eurométropole de Strasbourg, des engagements contractuels de l'État relatifs à l'autoroute A355. La commission a souhaité préciser et compléter ces dispositions, notamment le régime de sanctions, en le renforçant en cas de non-respect de l'interdiction du transit En définitive, le texte, tel qu'il a été enrichi par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et par la commission des lois, pour lequel je tiens à remercier le rapporteur pour avis

et l'Eurométropole de Strasbourg dans la mise en oeuvre des nouvelles compétences qui leur ont été attribuées, et de renforcer l'efficacité des dispositions initialement prévues dans les ordonnances. La commission a souhaité être à l'écoute des territoires concernés et relayer leurs préoccupations. C'est cette démarche qui a irrigué les orientations qu'elle a adoptées. La parole

l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de nous prononcer sur ce dispositif d'ordonnances, dont la ratification expresse par le Parlement n'est que trop rare, hélas. Toutefois, monsieur le ministre,

Notre assemblée a d'ailleurs pu se prononcer sur ce sujet dans le cadre de l'examen de l'excellente proposition de loi constitutionnelle déposée par notre

Ce préalable étant posé, je voudrais brièvement évoquer devant vous, mes chers collègues, les apports que la commission des lois a proposés sur ces trois ordonnances.

Les vingt amendements proposés par la commission et adoptés- souvent au bénéfice d'amendements déposés en des termes identiques par mon collègue Jean-Claude Anglars -visaient trois objectifs. Premièrement, nous avons cherché à assurer à la CEA des marges d'adaptation aux réalités locales, en garantissant, d'une part, la libre administration de l'institution, et, d'autre part, un accompagnement adéquat des services de l'État dans la mise en oeuvre du dispositif. Deuxièmement, notre travail fut de bâtir une taxe modèle, transposable, à l'avenir, aux collectivités territoriales volontaires- j'insiste sur ce dernier mot, dont je sais combien il tient à coeur

à l'échelle nationale, afin d'éviter à l'avenir toute disparité en la matière entre les collectivités territoriales qui mettraient en oeuvre ce dispositif.

de risques contentieux pour les collectivités concernées, et une norme nationale serait, en l'espèce, protectrice. Troisièmement, le dernier axe de notre travail, peut-être le plus essentiel à mes yeux, fut de garantir l'effectivité des contrôles et sanctions relatifs à la taxe, pour en assurer un meilleur rendement. C'est dans ce cadre que nous avons nous avons souhaité renforcer les moyens de contrôle, tout en les encadrant, simplifier les procédures et rétablir la proportionnalité des sanctions encourues. Si je me félicite que de nombreux ajouts n'ont pas fait l'objet d'amendements de suppression de la part du Gouvernement, je ne puis que regretter que, sur ce dernier volet, le Gouvernement souhaite revenir sur plusieurs dispositifs proposés par la commission. Il en est ainsi de la procédure de régularisation sans pénalité pour les redevables occasionnels, de la procédure de transaction, ou de la faculté d'installer, notamment pour les forces de l'ordre, des dispositifs de contrôle automatisés de la taxe.

le plus souvent à ouvrir des facultés aux collectivités territoriales. Ces apports me semblent consolider le dispositif de taxation et garantir le principe de la libre administration. Il s'agit donc plus que d'une occasion à saisir : c'est une nécessité, et je vous proposerai, mes chers collègues, de rejeter les amendements du Gouvernement en la matière. Je terminerai mon propos en saluant le rapporteur au fond de ce projet de loi, Jean-Claude Anglars, les qualités d'écoute ont permis un véritable travail commun de grande qualité. Le texte issu de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable nous satisfait sur l'ensemble des points dont la commission des lois s'était saisie saisie pour avis. Ce texte équilibré nous paraît à même de répondre à nos préoccupations partagées en faveur de la mobilité sur nos territoires. Nous passons

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à titre personnel, je suis favorable à ce projet de loi, et je tiens d'ailleurs à féliciter nos collègues parlementaires alsaciens pour n'ont pas baissé les bras devant l'adversité, et je leur souhaite que ce texte puisse aboutir de manière concrète. Si j'ai déposé cette motion, c'est parce que je voulais revenir sur la raison pour laquelle nous sommes ici à débattre de ce texte. Si nous sommes ici, c'est parce que l'excellente loi qui avait été votée à l'époque du président Sarkozy, avec l'accord et le soutien de tous les parlementaires, sur toutes les travées - ce texte faisait l'unanimité

ce ne sont pas seulement les « bonnets rouges » bretons. Ce sont surtout les parlementaires qui ont fait de la surenchère politicienne, à l'époque, en pourrissant

le dire beaucoup plus fermement et le déplorer beaucoup plus clairement dans le rapport de la commission, car il y a eu de l'irresponsabilité

au niveau national. Ils auront montré qu'il est possible de mettre en oeuvre une taxe sur le transit des poids lourds partout où c'est nécessaire. Quel

Les ajouts de la commission encadrent davantage les dispositions contenues dans les ordonnances. C'était nécessaire dans plusieurs cas précis, certaines des dispositions prises pour la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) pouvant à terme être dupliquées sur d'autres territoires, à des degrés différents. Je pense évidemment à la question de l'écotaxe, coeur névralgique du texte. C'est en tout cas le point qui a soulevé le plus d'interrogations, de modifications et de recherches de solutions.

Les conséquences seraient des pollutions sonores, mais également des pollutions de l'air et de l'environnement résultant d'un probable et problématique engorgement routier. Ce sera sûrement le cas du sillon mosellan.

de l'article 1 , qui prévoit une évaluation des reports de trafic sur les territoires voisins à la suite de la mise en oeuvre de l'écotaxe au sein de la CEA. Cependant, je m'interroge sur les mesures qui seront prises en conséquence.

Nous avons déjà dégagé les points positifs, et nous pourrons appréhender facilement les conséquences négatives. Il faudra toutefois faire attention à ne pas déplacer infiniment le problème. C'est pour cela qu'une coordination nationale et européenne devrait être engagée dans le même sens de ce qui a été fait sur la directive Eurovignette. Je me félicite d'ailleurs que la nouvelle version de cette dernière, censée entrer en vigueur dès 2023, soit prise en compte dans ce projet de loi.

D'une manière générale, les trois ordonnances proposent un rythme d'organisation cohérent concernant la compétence des routes et des autoroutes que récupère la CEA. L'exercice nous rappelle que la subsidiarité, la décentralisation et les relations entre États et collectivités territoriales sont indispensables et que les questions autoroutières n'ont pas fini de nous remuer les méninges. Nous serons vigilants et nous surveillerons avec une attention particulière l'application de ces textes.

resituer dans un contexte plus global. Ce projet de loi de ratification d'ordonnances, dont le point central est l'instauration de contributions face au trafic routier de marchandises, arrive quelques mois après l'examen de la loi Climat et résilience.

Ce texte est d'abord est une étape de vérité : la vérité des avis exprimés, des craintes ressenties. Le droit à l'alternative doit avoir le mérite d'exister.

Je veux tout d'abord parler de la crainte d'un report de trafic, ainsi que des difficultés créées en termes d'interopérabilité des systèmes. Je veux ensuite parler de la crainte de duplication d'un tel dispositif dans des régions où le transport de marchandises est un déterminant économique majeur. Je veux enfin parler de la position défendue par les territoires limitrophes, refusant d'être spectateurs des décisions de la Collectivité européenne d'Alsace. Voilà des inquiétudes pour lesquelles on ne saurait passer outre, sous peine de voir surgir une légitime levée de boucliers. Sur la base de ce travail de longue haleine, nous avons cherché le meilleur compromis possible tout en restant fidèles aux principes d'acceptabilité des mesures et d'effectivité sur le terrain, qui nous ont toujours guidés au Sénat et qui font l'honneur de la Haute Assemblée.

Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Cette solution a été partagée par tous mes collègues voilà maintenant quatre mois. Nous pouvons nous réjouir qu'elle conditionne le présent texte. En effet, nous nous sommes entendus, et cette position partagée a mené les excellents rapporteurs Jean-Claude Anglars et Stéphane Le Rudulier à décliner les modalités de la concertation. Désormais, le texte prévoit un cadre institutionnel favorisant la concertation de toutes les parties prenantes limitrophes de la Collectivité européenne d'Alsace, par l'intermédiaire d'un comité en amont

Personne ici- je l'imagine -ne conteste la faculté accordée à la Collectivité européenne d'Alsace de mettre en place le dispositif prévu. Personne ici- j'en suis certain -n'a oublié le cheminement qui a conduit à l'octroi de cette faculté, notamment la situation du report de trafic de l'Allemagne vers l'Alsace.

L'amendement de nos rapporteurs ne fait donc que se calquer sur ce que le Sénat a voté voilà quelques mois, en introduisant une concertation pour associer les territoires, notamment ceux de la région Grand Est. région Grand Est. Je ne m'étendrai pas sur les articles 2 et 5, dont les enjeux politiques sont manifestement moins prégnants. Selon moi, l'article qui met en place la concertation reste le plus important, tant il conditionne le mécanisme prévu tout en redonnant aux collectivités territoriales le pouvoir qui leur est dû. Je veux donc à ce stade féliciter sincèrement le rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Jean-Claude Anglars,

et résilience laissent transparaître un enjeu plus global que la seule taxation comme réponse unique à la transition écologique. Je me dois de vous rappeler, mes chers collègues, que nous ne saurions nous contenter d'une échelle seulement punitive sur la voie de la décarbonation des transports de marchandises. Instaurer une écotaxe ou une taxe poids lourds, aussi tentant ou nécessaire que cela puisse paraître, ne doit pas être une fin en soi. Nous avons toujours prôné une transition juste faisant de l'accompagnement et du soutien à la décarbonation un vecteur plus vertueux du changement de paradigme sur le transport. un chemin bien plus difficile, qui nous détourne de la voie plus aisée de la taxation. Mais il a le mérite de rendre plus acceptable la transition du secteur routier vers un modèle plus vert, désormais possible- j'y tiens tout particulièrement -l'utilisation du fret ferroviaire et du fret fluvial, pour lesquels nous avons désormais de grandes ambitions dans notre pays. Cette mise en perspective étant faite, la route est désormais tracée. Il ne nous reste qu'à nous y tenir. La parole

Il est temps ! Depuis une vingtaine d'années, le bassin rhénan est marqué par un total déséquilibre, dont pâtit lourdement la dorsale routière d'Alsace. Alors que les Suisses ont leur redevance poids lourds depuis 2001 et que les Allemands ont leur depuis 2005, notre pays n'a pas de dispositif similaire. L'Alsace,

Ainsi, au droit de Strasbourg, ce sont près de 14 000 poids lourds qui aggravent chaque jour les dégâts : congestion, pollution, atteintes à la santé, nuisances sonores, dégradation forte de la voirie, insécurité routière, concurrence faussée plombant toute chance de développement au fret ferroviaire ... Le contraste est accablant avec nos voisins européens de l'autre rive, qui ont su, eux, actionner le principe « pollueur-payeur », permettant de maîtriser mieux le flux de poids lourds, d'optimiser les charges transportées, de réduire les nuisances et d'assurer un fret ferroviaire significatif. Leur logistique s'est modernisée, et sa performance économique s'est améliorée. Les résultats avérés de ces politiques en font des pionnières en Europe. Le fret ferroviaire allemand est quatre fois plus important que le nôtre. L'effet de bord est massif, et c'est l'Alsace qui déguste : l'Alsace désarmée Il y a eu des tentatives pour réagir. Je pense à la bonne intention de la loi de 2006, arrachée par les élus d'Alsace, mais sans cesse décalée, sabotée, avant d'être balayée. Il y a eu l'ambition de l'écotaxe issue du Grenelle de l'environnement, ambition qui s'est fracassée de la manière que l'on sait Ce qu'en ont- hélas ! -retenu nombre de nos concitoyens d'Alsace, c'est l'incapacité des politiques publiques, la procrastination chronique et les renoncements successifs. Il faut en prendre la mesure : ces files continues de camions alimentent la déception populaire vis-à-vis d'une Europe qui n'arrive pas à réguler dans la cohésion, ainsi que la perte de confiance dans les capacités de notre démocratie à entendre les citoyens, à décider et à mettre en oeuvre. Il est donc temps d'entendre les citoyens et de ne plus laisser l'Alsace désarmée. C'était la volonté inscrite dans la loi instituant la CEA.

de ses délibérations précisant les tonnages, les catégories, le réseau taxable, les dispositifs technologiques retenus, les taux kilométriques, les majorations pour coûts externes, les réductions, les exonérations ... Il reste ainsi beaucoup à accomplir. L'entrée en vigueur ne sera pas

n'être pas à la hauteur des enjeux et des attentes. En l'occurrence, deux impératifs devraient servir de guides. Premièrement, la taxe alsacienne doit être d'un niveau équivalent à celui de la taxe allemande. Si elle devait viser clairement plus bas, nous aurions largement échoué à juguler les reports frontaliers. Deuxièmement, il ne faut plus perdre de temps ni retomber dans les travers qui ont tué la loi d'expérimentation régionale de 2006,

Ce délai maximum pour l'entrée en vigueur risque de jouer comme une incitation à décaler, à reporter, à déresponsabiliser avec le temps les nouveaux conseillers d'Alsace, qui ont pourtant été institués en premier lieu pour cette compétence et ce mandat explicites. Voilà pourquoi nous proposons de ramener ce délai à trois ans. de cet ordre qui a été annoncée à nos concitoyens par l'exécutif de la Collectivité européenne d'Alsace. Pour gagner efficacité et crédibilité, il s'agit faire au mieux sans traîner dans ce créneau. La mise en place de la taxe en Alsace a d'autant plus besoin d'un rythme fiable qu'elle est appelée à précéder une perspective similaire

Il y aura des effets de bord à prendre en compte. On entend l'inquiétude des riverains de l'autre dorsale routière, de l'autre côté des Vosges. Il y a des transitions différenciées, des imbrications délicates à préparer, une évolution à anticiper du droit européen. Mais faut-il que toutes ces difficultés soient des prétextes à l'immobilité ?

nous sommes donc invités à émettre un avis sur les ordonnances gouvernementales visant à permettre d'instaurer une écotaxe régionalisée en Alsace.

nous considérons que le projet pose des questions fondamentales sur lesquelles il n'est pas superflu de s'attarder. En effet, si l'on peut comprendre que les collectivités qui subissent quotidiennement les nuisances découlant de la circulation d'un trop grand nombre de camions, il n'en reste pas moins que toutes les régions de France ne sont pas confrontées aux mêmes réalités ni aux mêmes dynamiques économiques

a, si j'ose dire, la France. Eh oui ! Dès lors, une question fondamentale se pose. Devons-nous soutenir une décentralisation dans la République ou une décentralisation de la République ?

Il faut bien le reconnaître, les auditions que nous avons eues depuis lors ne nous rassurent pas totalement. Nous avons d'ailleurs constaté déjà qu'un certain nombre de réserves s'exprimaient sur le sujet.

incombe aux régions dans l'hypothèse où les collectivités de base ne l'assumeraient pas. Cela revient à dire que les régions auront à faire tout ce que les autres ne font pas. On appelle cela gérer les restes ; ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Une telle ambivalence- à tout le moins ! -n'est pas saine et risque de devenir très vite un sujet de controverses, voire de conflits entre différents échelons de collectivités. Si l'on y ajoute le fait que, en matière d'infrastructures routières, ce sont les départements qui restent les référents, il apparaît que nos lois récentes ont créé une forme d'incohérence dont nous pouvons déjà mesurer quelques effets compliqués.

Ainsi, les ressources financières qui résulteraient de l'instauration d'écotaxes régionales risqueraient d'aller alimenter les budgets généraux des collectivités, peut-être même pour entretenir les routes.

N'est pas levé enfin l'obstacle réglementaire européen qui, au nom de la concurrence « libre et non faussée », interdit de taxer les poids lourds étrangers et autres véhicules terrestres circulant en France. Il y a donc un risque très vraisemblable de taxation de tous camions, y compris de ceux qui assurent des trafics domestiques.

au sein duquel une régionalisation véritable pourrait trouver sa place. Ce sont autant de raisons qui nous conduisent à ne pas voter en faveur de la ratification

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la « naissance » que nous avons actée voilà deux ans maintenant de la Collectivité européenne d'Alsace et de ses compétences allouées, avec le transfert des routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national, nous permet aujourd'hui d'examiner une question particulièrement attendue en Alsace : la mise en place d'une taxe poids lourds. Ce sont en effet désormais la CEA et l'Eurométropole de Strasbourg qui gèrent et exploitent sur leurs territoires respectifs ces routes et autoroutes non concédées. Auparavant, cela relevait de l'État.

ans que notre territoire alsacien subit mécaniquement un report important du trafic poids lourds sur l'axe nord-sud, l'A35, depuis la mise en place d'une taxe poids lourds sur l'A5 allemande le 1 janvier 2005. Depuis cette date, ce sont des camions venus de toute l'Europe qui empruntent notre parallèle française gratuite et qui passent par Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Résultat, l'Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, assortie d'une paralysie élevée à certaines heures qui se traduit par voie de conséquence par une accidentologie élevée, sans parler des effets délétères en termes de santé publique, en raison de la forte augmentation de la pollution de l'air et du bruit. Lassé de voir les reports de poids lourds d'Allemagne- comme cela a été indiqué, il y a plus de 3 500 poids lourds supplémentaires par jour -sur les axes alsaciens, Adrien Zeller avait déjà multiplié les démarches voilà vingt ans pour appuyer l'instauration d'un tel dispositif sur notre territoire. Il plaidait pour une expérimentation en Alsace, avant une généralisation dans le reste du pays. En 2005, notre collègue, le député Yves Bur avait bien tenté de proposer une solution, avec la création d'une taxe poids lourds en Alsace. Cela avait d'ailleurs nourri les velléités de création d'une écotaxe nationale, option abandonnée en 2013 à la suite de la contestation des « bonnets rouges Une première loi avait d'ailleurs été votée dans les conditions que l'on sait : la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, instituant cette taxe à titre expérimental. Elle a par la suite connu de nombreux revirements. On se souvient à cet égard de la gabegie financière prévalant sous d'autres majorités, qui avaient remis en cause la taxe alors que les portiques visant à identifier les poids lourds avaient déjà été installés ; cela avait été fortement coûteux. Je me réjouis donc de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui et j'apporte bien évidemment mon entier soutien au projet de loi de ratification, qui représente un premier test susceptible d'être généralisé aux régions volontaires avec la loi de décentralisation en cours de discussion. Je salue à cet égard les travaux des commissions saisies, ainsi que des rapporteurs, sur l'ensemble du périmètre que sous-tend la mise en oeuvre de cette écotaxe. écotaxe. Ils ont su en adapter par voie d'amendements les modalités pratiques. Ce soutien n'est cependant pas exclusif de certaines problématiques qui ne manqueront pas d'alimenter durement les débats. Je pense notamment aux transporteurs locaux français, qui seront fortement pénalisés, mais également aux reports vers des axes secondaires gratuits, qui auront naturellement et inexorablement lieu. Sur le premier point, malgré un champ d'action particulièrement mince eu égard aux dispositions européennes, qui n'autorisent pas de différence de traitement entre les transporteurs en fonction de leur nationalité, de quelle marge de manoeuvre disposons-nous en termes de dérogations et/ou de compensations, afin de ne pas dégrader plus avant leur situation économique, leur compétitivité et, en bout de chaîne- nous le savons -, les finances des consommateurs ? Des systèmes peuvent être mis en place. Je pense par exemple aux modalités de remboursement ou de compensation en faveur des transporteurs nationaux. Sur le second point- je fais référence au report sur le réseau secondaire du trafic des poids lourds qui choisissent d'éviter les autoroutes à péage -, nos travaux de qualité au Sénat ont permis de dégager des solutions pragmatiques qu'il serait judicieux de mettre en oeuvre sans délai. Le récent rapport que mes collègues Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau ont remis au nom de la commission du développement durable a en effet parfaitement restitué les tenants et aboutissants d'un tel phénomène, ainsi que les moyens de lutter contre ses externalités négatives cartographier les principaux « itinéraires de fuite » et permettre aux élus locaux d'actionner des leviers de réduction des nuisances de manière différenciée, agir sur les motorisations du parc de poids lourds en permettant un « verdissement » efficace et dépasser les divergences actuelles, équilibrer la fiscalité du transport de marchandises en définissant un cadre national harmonisé et prenant en compte une tarification kilométrique, appliquée avec pragmatisme. Traiter de manière pragmatique l'ensemble des situations qui vont découler de la mise en place de cette taxation des poids lourds est la condition de son acceptabilité et de son efficacité.

la ratification de ces ordonnances, qui représentent une avancée importante à l'heure de la COP26 et des préoccupations de nos citoyens relativement au changement climatique. Je voudrais également saluer le travail remarquable des deux rapporteurs, Jean-Claude Anglars et Stéphane Le Rudulier. Mes chers